la parole sera donnée à l'auteur du débat, à un orateur de chaque groupe, puis aux ministres pour leur répondre. Ensuite, nous procéderons à une séquence de seize questions-réponses.

Le Sénat- j'en suis convaincu -s'honore de ce moment de vie parlementaire et démocratique. Il est exceptionnel, aussi bien par sa forme, qui prévoit un temps d'expression réservé aux groupes politiques, que par le sujet traité, l'opération Barkhane. Je voudrais également vous remercier, monsieur le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, madame la ministre des armées, d'avoir bien voulu participer à ce débat. Loin de tout esprit politique,

il est sans doute bon que les institutions jouent leur rôle en permettant une expression diverse mais constructive. Ce débat est d'abord l'occasion de saluer une fois encore l'engagement exceptionnelde nos militaires.

Nous nous inclinons devant leur mémoire. Notre reconnaissance et notre soutien vont bien sûr aussi aux nombreux blessés. Nous ne les oublions pas Expliquer leur action et le sens de leur mission, comme nous allons le faire cet après-midi, est sans doute la meilleure manière de leur rendre hommage. Le 22 avril 2013, nous avons autorisé la prolongation de l'opération Serval, conformément à l'article 35 de la Constitution. Près de huit ans plus tard, Serval est devenue Barkhane, et la France est toujours engagée au Sahel. En huit ans, les modalités de notre engagement ont beaucoup évolué.

L'État islamique dans le Grand Sahara est monté en puissance : les attaques djihadistes se sont étendues dans le centre du Mali, dans la zone des trois frontières puis au Burkina Faso, et menacent maintenant tout le golfe de Guinée. Quelques jours avant le sommet de N'Djamena, il est donc temps de faire ensemble le point sur cet engagement de longue haleine et de tracer de nouvelles perspectives. À cet égard, savoir si 600 soldats vont ou non quitter Barkhane est certes important, mais n'apporte pas totalement la réponse que nous attendons. Nous souhaitons avant tout comprendre la stratégie du Gouvernement pour la période à venir.

nous sommes parvenus à mobiliser le soutien d'un certain nombre d'alliés européens, même si les moyens qu'ils ont mis en oeuvre nous paraissent encore insuffisants. La force Takuba a pu commencer à entrer en action. Les armées de nos alliés du G5 Sahel ont également progressé, souvent en payant le prix du sang. Nous devons leur rendre hommage, car le tribut qu'ils ont payé est indiscutablement un prix très fort dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, grâce à la pression exercée en permanence par nos forces et par celles de nos alliés, la constitution d'un sanctuaire djihadiste a pu être évitée, ce qui était l'objectif initial. Un autre constat, cependant, s'impose à nous : le dénouement de cette crise, qui dure depuis huit ans, ne sera certainement pas militaire, nous le savons. La solution ne peut être que politique. Par conséquent, elle est essentiellement du ressort des Maliens eux-mêmes. Or les accords d'Alger n'ont pas été appliqués. Pis, le nouveau coup d'État au Mali nous donne parfois l'impression d'un retour en arrière de près de huit ans. Dans ces conditions, allons-nous signer pour un nouveau bail de huit ans ? Que se passera-t-il si, au terme de cette période, rien n'a changé sur le plan politique au Mali ? Mali ? Nous ne pensons pas qu'un retrait brutal de nos armées soit la bonne réponse ; ce ne serait ni conforme à nos intérêts ni à celui de nos alliés qui ont demandé notre aide. Nos choix doivent consolider les acquis de Barkhane, et non les sacrifier. Mais nous sommes en droit, compte tenu de notre engagement et du prix que nous payons, d'attendre des progrès sur la voie de la réconciliation nationale malienne.

Les Français veulent tout simplement savoir quel est le plan du Gouvernement pour qu'un jour la France puisse retirer ses forces sans craindre un nouveau séisme. De notre côté, nos travaux ont mis en évidence le caractère crucial du développement économique et, par conséquent, celui de l'aide publique au développement. C'est essentiel pour lutter contre les causes profondes du terrorisme au Sahel. Sans cela, nous ne traiterons que les symptômes, et les populations locales finiront par nous voir comme des troupes d'occupation. Nous avons dépensé 900 millions d'euros pour Barkhane en 2019, contre seulement 85 millions d'euros en aide publique au développement nette pour le Mali. Certes, nous ne sommes pas seuls : l'Alliance Sahel, créée en 2017, a également mobilisé des sommes très importantes. Toutefois, il nous reste très difficile d'atteindre des régions qui en ont le plus besoin, particulièrement au nord du Mali. C'est pourtant la seule façon d'offrir des perspectives aux jeunes de ces territoires. Éducation, santé, services publics de base : telles sont les améliorations concrètes que les populations attendent et qu'elles doivent voir enfin arriver. La future loi d'orientation sur la solidarité internationale, que nous allons enfin pouvoir examiner dans quelques semaines, sera l'occasion de réorienter encore davantage Enfin, notre débat d'aujourd'hui doit être l'occasion d'aborder des préoccupations plus immédiates. La protection de nos soldats constitue pour nous une priorité absolue. Qu'en est-il du renforcement du blindage des véhicules légers que nous attendons encore ? Ne faut-il pas basculer dans la mesure du possible vers davantage d'aéromobilité, puisque les principaux attentats qui touchent nos troupes interviennent à l'occasion de convois automobiles ? de convois automobiles ? À cet égard, j'ose croire que l'actualisation de la loi de programmation militaire nous permettra aussi d'aborder directement ce sujet. vous l'aurez compris, nous sommes loin de toute posture. La diversité des points de vue qui vont s'exprimer le montrera. Nous sommes face à une situation difficile, complexe. Il n'y a pas de solution toute faite, mais nous devons nous confronter ensemble à cette complexité. Tel est le rôle du Parlement. Mes chers collègues, ce débat est aussi un symbole. Il s'adresse à nos concitoyens pour qu'ils sachent que, partout où la France se bat, c'est pour faire progresser la paix. Quant à nos soldats qui patrouillent en ce moment même dans les déserts brûlants et dangereux du Sahel, puissent-ils accueillir ce débat comme la marque de notre confiance et de notre soutien. Ils sont la fierté de la France

à ces femmes et à ces hommes d'exception engagés au Sahel, dont la combativité et le dévouement sont inégalables. Leur abnégation est un modèle pour nous tous. Je veux leur dire, au nom du groupe RDPI, combien nous sommes fiers d'eux et combien nous leur sommes reconnaissants. Ils peuvent compter sur notre soutien indéfectible. À tous nos soldats tombés au service de notre nation, je rends également un hommage ému et sincère. La tenue de ce débat tombe à point nommé, puisqu'il se déroule à quelques jours d'un sommet déterminant à N'Djamena. Il nous donne l'occasion de réaffirmer l'action capitale que mène la force Barkhane et de renouveler toute notre confiance au Président de la République et à son gouvernement. Les groupes armés terroristes que nos soldats combattent, hier avec l'opération Serval pour les empêcher de provoquer la chute d'un État allié, le Mali, et aujourd'hui avec Barkhane pour les empêcher de faire de la bande sahélo-saharienne une base arrière du terrorisme de la taille de l'Europe, représentent une menace bien tangible. Mais, en passant de Serval à Barkhane, nous sommes passés d'une guerre d'intervention courte et rapide à une guerre d'un tout autre genre. Nous avons pleinement conscience que, sans nos soldats sur place, aux côtés des armées sahéliennes, cette menace s'étendra demain à toute l'Afrique de l'Ouest. C'est parce que nos partenaires européens partagent pleinement cette analyse qu'ils s'investissent chaque jour un peu plus au Sahel. Cela me donne l'occasion de saluer l'engagement de nos alliés européens, que ce soit au sein de la Takuba ou dans d'autres opérations. Depuis le sommet de Pau, Barkhane a fortement accéléré le rythme de neutralisation des groupes terroristes. la montée en puissance des forces sahéliennes est encourageante, bien que celles-ci ne soient toujours pas en mesure de prendre la relève intégrale de Barkhane et d'affronter seules la menace des groupes armés. Au côté du rôle essentiel de la France, une addition de faiblesses ne fait pas une force. Si nos armées remportent chaque jour des victoires tactiques, il nous faut prendre conscience que la crise est aussi politique et économique. Comme il est stipulé dans les quatre piliers complémentaires du sommet de Pau, nous devons transformer ensemble les gains durement acquis sur le terrain en progrès politiques, économiques et sociaux et trouver un moyen de sortir l'approche « 3D »- diplomatie, défense, développement -de sa phase incantatoire. faire, nous avons besoin d'engagements forts de la part de nos partenaires sahéliens, surtout maliens. Il faut une feuille de route claire en faveur d'une bonne gouvernance politique démocratique et du développement de services publics dans les zones fragiles- je pense notamment aux zones du Nord Nord -, nécessaires pour restaurer la confiance en l'État, de la tenue d'élections en mars 2022, de la préservation de l'espace humanitaire et du développement de nouveaux ponts économiques, de la lutte contre la corruption, les trafics humains, de stupéfiants et de produits de contrebande en tout genre, qui gangrènent la société et favorisent l'insécurité et l'instabilité.

Du racisme à rebours à l'anticolonialisme primaire, en passant par la réécriture de l'Histoire, leur caractéristique commune est le dénigrement de l'action passée, présente et future de notre pays en Afrique. Nous le voyons bien, en parallèle du cadre strictement militaire, il existe toute une série d'autres combats à mener, qui prennent beaucoup de temps et qu'il s'agit de concrétiser rapidement sous peine d'enlisement.

Monsieur le ministre, par quels moyens politiques et diplomatiques envisagez-vous d'intervenir pour assurer la mise en oeuvre concrète de cet accord de paix ? Avec quels acteurs comptez-vous avancer et dialoguer, alors que le paysage régional comprend une myriade de protagonistes locaux armés ayant leurs propres agendas locaux ? Comment lutter contre l'instrumentalisation malveillante des opinions publiques locales et la propagation de fausses informations à des fins de politique intérieure ou par des puissances étrangères qui sapent nos efforts communs ? Le temps joue contre nous. C'est malheureusement une règle universelle : plus une opération militaire dure, plus la population locale a tendance à attribuer aux soldats la responsabilité de certaines situations. Pacifier ces pays en faisant naître un réel sentiment d'appartenance nationale passera par le développement. Tous ces objectifs ne pourront être atteints sans l'aide de la France et des acteurs étatiques et économiques sur place. La parole

À un an de l'élection présidentielle française, à quelques jours du sommet du G5 Sahel à N'Djamena, ne comptez pas sur moi pour polémiquer sur un dossier qui engage la France. La présence de 5 100 enfants de la Nation sur ce territoire sahélo-saharien appelle à des échanges responsables, loin des querelles politiciennes.

Je ne vais pas distribuer les bons ou les mauvais points de ce choix stratégique et géopolitique. En revanche, je tiens à poser les enjeux actuels de cette opération, qui s'éternise malheureusement. peut-elle pour autant justifier un retrait, voire une réduction de notre niveau d'engagement, alors même qu'António Guterres insiste dans son rapport trimestriel relatif à la situation au Mali sur le degré de violence auquel est confrontée la population ? Rappelons tout de même les raisons de notre présence au Mali à la demande du gouvernement de ce pays. Barkhane, c'est un gage de stabilité dans une zone en souffrance, un besoin réel pour contenir le terrorisme et ses nombreuses répercussions en Europe et sur notre territoire, un engagement à la formation de militaires maliens, un projet « araignée » d'aide à la population, une influence de la France. À l'occasion de ses voeux aux armées, Emmanuel Macron a rappelé que, « face aux risques de destruction des relations internationales et de notre société, les armées françaises ont été un facteur de stabilité, de force et de résistance ». Barkhane est entièrement résumée dans cette phrase. Notre présence a pour objectif de garantir une sécurité pérenne sur ce territoire, en partenariat avec les forces de Bamako et du G5 Sahel. La zone des trois frontières, à cheval entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est l'un des poumons des troupes djihadistes, aujourd'hui réunies sous la bannière de l'État islamique dans le Grand Sahara, branche locale de l'EI. L'enjeu est bel et bien de contenir le terrorisme, dont nous mesurons, hélas ! les répercussions en France et en Europe. Barkhane, c'est certes une présence militaire, mais ce sont aussi des projets d'aide à la population tendant à faciliter l'accès à l'eau, à l'énergie, à la santé, aux médicaments gratuits. Ils sont destinés à accompagner la population plutôt que de la laisser traverser la Méditerranée dans des conditions inhumaines. sont sans doute insuffisants- j'en conviens -, mais ils sont indispensables. L'avenir de ces populations n'est pas dans la migration, mais bien dans le développement du Mali et de la bande sahélo-saharienne. C'est pourquoi Barkhane est également un engagement à la formation de militaires maliens, fondement de la lutte active contre le terrorisme qui ronge ce territoire en terrorisant la population. Pérenniser notre intervention, si durable soit-elle, si douloureuse soit-elle, si chère soit-elle, demeure un enjeu géostratégique, un enjeu de coopération, un enjeu humain. notre engagement est l'un des fondements de notre influence en Afrique et dans le monde. Oui, notre présence représente une dépense

Notre politique d'influence en matière de défense mérite mieux que des projections budgétaires contraintes et la crainte de pertes humaines parmi les militaires.

Jean-Marie Bockel, après la perte de son fils : « Nous sommes infiniment tristes et fiers aussi de notre enfant. C'était un soldat engagé qui savait pourquoi il était là. »

Il n'est plus acceptable de placer le Parlement devant le fait accompli alors que, dans quelques jours à N'Djamena, le Président de la République devrait annoncer une fois de plus d'importantes décisions. Madame la ministre, vous avez déclaré devant notre commission : « Dire que la France est engluée dans une guerre sans fin est faux. » De notre côté, nous pensons que rien ne serait plus faux que de ne pas interroger sans concession les résultats de l'opération Barkhane. Vous ne trouverez pas plus farouches opposants aux terroristes islamistes que les communistes. Les démocrates que nous soutenons à travers le monde sont partout pourchassés et tués par ces groupes. Nos combats émancipateurs sont menacés par leurs visées obscurantistes. huit années de guerre au Mali ont-ils éteint ou propagé le feu du terrorisme islamiste et de tous les entrepreneurs de violence ? Le Mali vit-il davantage en paix qu'il y a huit ans ? Poser ces questions, c'est malheureusement y répondre. De plus en plus de Maliens, les populations civiles des pays du Sahel, ainsi que des militaires, des diplomates, des universitaires français posent ces questions avec nous.

La situation humaine, politique et économique du Mali empire. Dans ce contexte de déstabilisation sociale et politique, les islamistes continuent de développer leur sinistre entreprise. Les leçons des guerres menées au nom de la « guerre contre le terrorisme » ne sont pas tirées. Chaque fois, les pays sont laissés en proie au chaos pour des décennies. La désintégration de la Libye en est un exemple. Elle est d'ailleurs directement à l'origine d'une partie des violences armées dans le nord du Mali. Dans quel état laisserons-nous le Mali et les autres pays de la région si nous poursuivons dans cette voie ? Censés venir pour protéger le Mali, nous jouons aux apprentis sorciers, réveillant les divisions pour trouver des alliés, prétendant choisir entre les bons et les mauvais groupes armés, nourrissant la relance des conflits communautaires, jouant un jeu trouble avec le Mouvement national de libération de l'Azawad, suscitant la défiance des Maliens devant le risque d'une partition du pays qu'entérinerait la mainmise de groupes armés islamistes ou non sur le Nord. C'est d'ailleurs pourquoi les accords d'Alger ne peuvent être invoqués comme « la » solution politique et doivent être profondément révisés. Les islamistes prospèrent sur ces divisions, recrutent en exploitant le désespoir de populations spoliées de toute part. Nous devons tirer les leçons et tourner la page de Barkhane, car l'impasse est certaine. Il faut créer les conditions d'un départ programmé de nos troupes, de lui substituer un nouvel agenda politique, économique et de sécurité pour le Mali et la région. Cela ne se fera pas en un jour, car le mal est fait. Il ne s'agit évidemment pas d'abandonner le Mali au chaos.

Notre appui militaire doit être recentré sur le soutien aux armées locales, en retenant la formule d'un comité d'état-major conjoint des forces africaines qui exclue les puissances étrangères. La France doit soutenir avec vigueur la feuille de route de Lusaka baptisée « Faire taire les armes en participer à toute initiative multilatérale visant le désarmement de tous les groupes armés non étatiques, ainsi- c'est très important -que la lutte contre les flux financiers illicites qui subventionnent les trafics, les violences et les guerres en Afrique. Mais, plus que tout, c'est notre agenda politique qui doit changer. La France et l'Union européenne doivent encourager par tous les moyens, et en priorité sur les territoires les plus délaissés par les pouvoirs publics, de vastes plans d'action pour le développement. Les populations africaines, et singulièrement leur jeunesse, ont les ressources pour le construire et les entretenir. Les pays africains doivent sortir de la domination et d'un modèle d'économie extravertie, tourné vers les besoins des multinationales et d'élites aisées corrompues, car c'est le mal profond dont nous sommes encore les complices. La France doit massivement augmenter son aide publique au développement en révisant ses objectifs. Notre pays doit agir sans tarder pour mettre à disposition de ces pays

une maîtrise locale des ressources et la valorisation de capacités productives propres. Tel est l'intérêt des Africains ; tel est aussi notre intérêt. Le développement ne doit pas rester le troisième « D »,

En effet, depuis neuf ans que nous avons débuté notre intervention au Mali et au Sahel, ce n'est que la seconde fois que nous avons l'occasion d'avoir un débat de fond sur la stratégie, les enjeux et les perspectives de l'opération Barkhane. Barkhane. Je tiens à saluer unanimement l'engagement opérationnel de nos forces mobilisées sur les différents théâtres d'opérations de cette bande sahélo-saharienne, au Mali comme au Niger. Sur ce territoire grand comme l'Europe tout entière et au climat des plus arides, nos militaires mènent une lutte sans relâche contre le terrorisme et le fanatisme, parfois au péril de leur vie. Je veux avoir une pensée pour nos soldats tombés au combat, leurs frères d'armes, leurs proches, leurs familles. Mes pensées vont également en cet instant à notre ami et ancien collègue Jean Marie Bockel. Les opérations Serval puis Barkhane ont permis d'empêcher l'installation d'un califat territorial au Mali et la création d'un sanctuaire djihadiste comparable à celui qu'a instauré Daech Cependant, malgré de nombreuses victoires stratégiques et la neutralisation de nombreux chefs de groupes armés terroristes, force est de constater que la guerre est loin d'être gagnée. L'histoire nous démontre que l'intervention de pays occidentaux sur des théâtres d'opérations extérieures s'apparente le plus souvent à des conflits asymétriques forces militaires conventionnelles, d'un côté, groupes armés terroristes noyés au sein des populations, de l'autre. Pourtant, cette asymétrie ne confère pas une supériorité très évidente et ne permet pas à nos forces de vaincre la détermination, l'imagination et la mobilité opérationnelle de ces groupes armés, qui évoluent en effectif réduit et sur un terrain qu'ils connaissent parfaitement. Force est aussi de constater que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, loin de s'être améliorée, s'est véritablement dégradée le conflit originel au nord du Mali s'est régionalisé ; il s'étend désormais vers le sud jusqu'au Burkina Faso et se propage jusqu'aux pays riverains du golfe de Guinée. Aux conflits interethniques plus locaux se mêlent désormais les revendications idéologiques et religieuses. Ainsi, les forces françaises apparaissent bien seules sur ce terrain. Depuis neuf ans, l'engouement des autres pays européens à s'engager aux côtés de la France demeure peu visible par l'opinion publique. Est-ce seulement parce que la France est encore l'une des seules nations européennes à disposer d'une armée d'emploi, madame la ministre ? Pourtant, la poursuite de notre engagement dans cette bande sahélo-saharienne nécessite indiscutablement une coopération européenne et internationale élargie et renforcée, ainsi qu'une prise de conscience de tous les États membres de l'Union de l'intérêt qu'il y a à lutter collectivement contre le terrorisme, au plus près de ses racines dans cette région du monde. Cette coopération européenne ne peut se limiter à la mission européenne de formation de l'armée malienne. Celle-ci s'inscrit certes dans une approche globale pour renforcer les capacités militaires en vue de garantir l'intégrité territoriale,

Ce dispositif nous paraît à ce jour insuffisant pour faire face à la progression vers le sud de la zone d'influence des groupes armés terroristes. Il doit rapidement s'étendre de façon effective à tous les États membres de la CEDEAO, que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo ou le Bénin. Il s'avère désormais indispensable d'associer plus largement les pays riverains du golfe de Guinée. Lors du sommet de Pau, les chefs d'État du G5 Sahel ont réaffirmé leur volonté de renforcer cette force conjointe. Son élargissement sera-t-il pour autant évoqué lors du prochain sommet de N'Djamena ? Lorsque l'on évoque la collaboration européenne, il faut également parler de la Takuba, que vous appelez de vos voeux, madame la ministre, pour soutenir l'opération Barkhane. Cette composante de forces spéciales était également censée matérialiser l'engagement de l'Europe et renforcer la logique d'un partenariat de combat. Au-delà des bonnes intentions de nos voisins, les premiers éléments des forces spéciales françaises et estoniennes sont arrivés sur le théâtre des opérations. Mais qu'en est-il de l'engagement de nos autres partenaires ? Pouvez-vous nous indiquer de façon précise, madame la ministre, comment s'effectuera la montée en puissance de Takuba ? Une stratégie qui repose sur les deux piliers que sont l'« européanisation » et la « sahélisation » sera-t-elle suffisante pour sortir du conflit ? La question reste posée. Sans les citer, nous ne pouvons ignorer les velléités de certains États puissances très intéressés par cette région du monde et, plus particulièrement, par le continent africain. Alors, certes, il n'y a pas de petites victoires dans une guerre à condition qu'il soit envisageable de la gagner. Celle que la France mène au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane avec ses alliés ne pourra se solder que par une implication politique plus forte, à commencer par celle des pays concernés. Nous sommes tous conscients que l'absence de l'État dans ses missions régaliennes, que ce soit l'administration publique, les services de santé, l'éducation ou l'accès à des besoins vitaux, ne peut que favoriser l'emprise de groupes armés terroristes sur les populations locales. difficile dans ces conditions de percevoir l'État comme protecteur et non comme prédateur. Sans un État plus fort, la paix sera impossible.

Même s'il n'est pas envisageable d'opérer une réduction massive de l'empreinte française sur le terrain, une réflexion sur un accompagnement à forte valeur ajoutée de notre participation- drones, renseignements ou frappes aériennes ciblées -ne doit pas être occultée. À l'heure actuelle, le besoin prioritaire est d'établir une stratégie claire et un calendrier de transition adapté aux forces en présence, car la situation en Afrique de l'Ouest demeure d'une grande complexité.

de N'Djamena devra bien entendu permettre de réaffirmer la volonté des pays du G5 Sahel, mais également de solliciter une véritable implication des pays qui sont désormais menacés. Ensuite, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a déclaré il y a quelques jours vouloir renouer avec le multilatéralisme et réinstaurer le dialogue avec l'Union africaine, afin « de faire face aux périls les plus imminents ». Mes chers collègues, l'issue de ce conflit sera politique ou ne sera pas. Réfléchissons à ce que disait Paul Valéry : « Les guerres, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent parce que d'autres qui se connaissent très bien ne parviennent pas à se mettre d'accord. » La parole est à M. Jean-Marc

intervention sans avoir à mon tour, au nom du groupe socialiste, une pensée pour nos militaires, leurs familles et leurs proches. À ce jour, plus de 5 000 militaires sont engagés dans l'opération Barkhane.

Alors secrétaire d'État à vos côtés, monsieur le ministre, je garde le souvenir de celles et de ceux que j'ai croisés, de leur professionnalisme indiscutable, de leur très haut niveau d'entraînement, de leur détermination sans faille, de leur courage en somme. Ce qui m'a frappé et qui restera gravé en moi, c'est que revient toujours dans les yeux et les mots des proches de celles et ceux qui sont morts au combat le sens du devoir. On entend chaque fois cette phrase : « Nous n'aurions jamais pu le ou la dissuader de partir en opération, d'être aux côtés de ses camarades pour servir. Dans un monde où l'on ne cesse d'observer les effets de l'individualisme, nos militaires, dont la plupart sont très jeunes, démentent les idées reçues. Ensemble, avec leurs familles et leurs proches, avec tous les Français aussi, ils ne font qu'un. Il est important de rappeler régulièrement engagement et de le mettre en valeur. Je ne reviendrai pas longuement sur les raisons qui ont conduit à la situation actuelle. Ces éléments sont connus. Loin des et des réseaux sociaux, l'opération Barkhane a été lancée le 1août 2014. Elle fait suite à l'opération Serval, mise en oeuvre à partir du 11 janvier 2013. Rappelons-nous toujours qu'en quelques heures, à l'appel du Président démocratiquement élu du Mali, François Hollande, Président de la République française, alors commandant en chef de nos armées, a dû prendre la difficile décision de recourir à l'usage de la force pour protéger la liberté à plus de 6 000 kilomètres de chez nous. est la seule raison de notre présence au Mali : la liberté. Nous serons toutes et tous d'accord ici, et par-delà nos travées, pour saluer le courage de cette décision, celle du Président François Hollande. La France s'est honorée de ne pas rester les bras croisés quand le peuple malien a fait appel à elle. Cette décision était nécessaire, responsable et digne. Dans les faits, cette première bataille a été remportée en quelques semaines. Dès les premières heures, le dispositif français se déployait, démontrant une fois de plus les exceptionnelles capacités opérationnelles de projection de de projection de l'ensemble de nos forces armées. Oui, la France fait partie d'un club mondial très fermé, celui des nations capables de projeter massivement leurs forces dans le cadre d'opérations extérieures Au nom de nos valeurs, ces capacités militaires exceptionnelles confèrent, dans le concert des nations, une responsabilité supplémentaire dont notre pays a pleinement conscience. Ces derniers temps, nous entendons et lisons des choses insupportables pour la raison, dénuées de tout fondement rationnel. Il est essentiel de rappeler régulièrement les faits, les causes et les objectifs, ne pas laisser s'installer des rumeurs nauséabondes pour notre pays, mais plus encore et plus largement pour la démocratie. La France n'est pas un pays impérialiste, colonisateur ou déstabilisateur. La France ne poursuit qu'un seul but : la paix d'abord et avant toute autre considération, la paix dans la dignité pour les peuples, la paix, ici, au Mali et dans les pays voisins, pour que les peuples de cette région aient la possibilité de vivre librement, sans être maintenus sous le joug quotidien du terrorisme et de son aboutissement politique, dont la communauté internationale sait ce qu'il représente pour les peuples afghan, irakien, syrien et tous les autres. Redire la véracité des faits n'a rien d'artificiel dans un contexte de développement de suspicions, notamment dans le pot-pourri qu'est de plus en plus souvent internet, où tout se mélange. Face aux attaques dans le cyberespace, dont nous savons qu'au moins deux grandes puissances n'hésitent plus à faire un usage assidu, la vérité des faits est essentielle. Il faut en effet toujours revenir aux causes profondes pour déterminer la situation telle qu'elle se présente. En ce sens, ne serait-il pas plus urgent d'associer régulièrement les parlementaires et, notamment, de leur donner plus de moyens, afin qu'ils exercent leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif, un pouvoir traditionnellement relégué au second plan sur ces questions sensibles Nous avons ici l'occasion de changer de prisme et d'améliorer nos pratiques pour ne pas laisser le poison des rumeurs se propager et en revenir à l'objectivité des faits. Si, tactiquement, le succès de nos opérations militaires est indiscutable, il est tout aussi essentiel de débattre de notre stratégie, comme nous le faisons aujourd'hui. En décembre 2015, le gouvernement,

Pour agir sereinement et efficacement, la nature de la réponse doit nous conduire à reposer régulièrement cette question. Cet ennemi est effectivement mouvant, en évolution permanente, immergé dans les sociétés pour déstabiliser les États et tenter d'y diffuser un ensemble idéologique à rebours de la liberté, perspective, ne l'oublions jamais, d'instauration de proto-États de type Daech. Cette situation ne relève ni des angoisses ni des fantasmes du monde occidental. C'est la réalité du terrain, telle qu'elle a été décrite, notamment, dans le Livre blanc de 2013. Pour faire face, la France n'a jamais eu la culture et l'obsession de la guerre préventive, là où d'autres pays ont pu s'y confondre, prenant le risque de s'y perdre moralement, culturellement et économiquement. Les comparaisons avec ces pays, si elles pourraient avoir le mérite de questionner notre stratégie- ce qui est nécessaire -, retomberaient immédiatement à l'épreuve des faits. la France, fidèle à ses valeurs et à sa tradition, a intégré que la sécurité absolue est un leurre et que l'ennemi doit sans cesse être redéfini, au plus juste et en réaction. Au Mali, comme ailleurs, notre stratégie ne varie pas : la France ne mène aucune guerre préventive ; la stratégie française est défensive et dissuasive. Je le disais, ce débat est nécessaire, parce qu'il faut toujours questionner et redéfinir l'ennemi au plus juste, parce qu'il s'agit, aussi, de dépasser le simple cadre militaire. Pour ne pas sombrer dans ce chaos où des forces obscures connues souhaitent entraîner les pays de la région, en premier lieu le Mali, y compris lorsqu'elles sont couronnées de succès, ne suffisent pas. Elles peuvent même conduire à l'impasse sans une approche globale politique, diplomatique, économique, éducative et judiciaire. Nous le savons, une stratégie durable repose sur cet éventail de dispositions. Or, madame la ministre, le sentiment grandissant, dans les médias, mais aussi, à bien des égards, sur le terrain opérationnel et parfois même jusque dans nos armées, c'est que ces dispositions, par-delà les opérations militaires, sont de moins en moins visibles. Madame la ministre, monsieur le ministre, vous le savez, de nombreuses questions sont posées. Je me permets d'en relayer quelques-unes. Où en sommes-nous sur le terrain diplomatique, notamment au sein du G5 Sahel ? Nous le savons, la situation en Libye est loin d'être stabilisée ; quels sont les effets de la crise libyenne pour la zone de travail de Barkhane ? Peut-on s'attendre à un changement d'attitude de la part des États-Unis et de la nouvelle administration du Président Biden ? Sans tomber dans le risque opérationnel que ferait courir la publication d'un calendrier, à quelle échéance les pays auront-ils localement suffisamment de moyens pour prendre le relais militaire ? En d'autres termes, où en sommes-nous de la formation et de l'accompagnement ? Dans les champs économique et éducatif, comment accompagnons-nous les pays menacés ? Quels sont les projets structurants qui permettront aux territoires du Nord, où la misère est grandissante, de sortir de l'impasse ?

a été confiée à notre armée : lutter contre les groupes armés terroristes. Elle l'a admirablement accomplie et continue de le faire. Nos soldats ont ainsi libéré les villes occupées et poursuivent les terroristes partout où ils se trouvent. Ce n'est pas au moment où le bilan de l'opération Barkhane s'améliore, alors que de nouveaux entrants européens viennent nous épauler, Le principal effet de l'opération Barkhane est de prévenir l'effondrement des États et la création d'un sanctuaire par les terroristes. Tout retrait donnerait satisfaction aux activistes qui sont, par nature, nos ennemis. Ne nous y trompons pas ! Les armées locales sont encore loin d'être en mesure de lutter seules contre ces groupes. Un retrait de nos forces serait suivi d'une nette dégradation des conditions de sécurité, qui entraînerait des déplacements massifs de population. Au coeur du Sahel, contrairement à la désinformation des réseaux sociaux, la population malienne, à une très forte majorité, aspire au maintien de la présence militaire française. Notre pays peut s'enorgueillir de son action. Le sacrifice de nos soldats pour une juste cause n'est pas vain. La tâche est considérable. Pour fonder une paix durable, les nations de la zone doivent renforcer leur unité. Les États et leurs services publics doivent également être capables d'assurer une présence auprès de toutes les populations et sur tous les territoires. J'illustrerai mes propos par l'exemple d'une ville que je connais bien. En 1995, j'ai initié une coopération décentralisée entre ma ville et celle de Kati, limitrophe de Bamako. Aujourd'hui, la situation y est catastrophique.

de 30 millions à 9 millions de francs CFA. Connaissez-vous beaucoup de villes pauvres qui pourraient supporter une baisse de 70 % de leur budget ? Les agents territoriaux ne sont plus rémunérés. À Bamako, il est de plus en plus difficile de circuler. La misère se développe, par manque de travail et de ressources alimentaires, mais aussi par l'arrivée de déplacés fuyant les zones dangereuses. Nos amis Maliens souffrent sur les plans économique, touristique, sécuritaire et politique. Sur le plan économique, les partenaires d'hier commencent à manquer cruellement. Les aidants sont de plus en plus rares. Sur le plan touristique, les villes de Ségou et de Mopti, qui connaissaient un flux régulier de touristes, ont perdu une ressource précieuse.

Cette situation est extrêmement grave, car c'est sur ce terreau que croît l'effervescence radicale terroriste. Aussi, sur le plan politique, les gouvernants des États du Sahel doivent affronter une situation très complexe. Les écoles doivent rouvrir. Pour affaiblir et faire disparaître les groupes armés terroristes, il faut agir à tous les niveaux. L'opération Barkhane ne saurait, à elle seule, résoudre le phénomène terroriste au Sahel. Elle est une condition nécessaire à l'émergence de solutions politiques. Si la zone passait sous le contrôle des terroristes, comme ce fut le cas en Afghanistan ou au Levant, le risque serait grand de voir la violence s'exporter contre nos populations. Nous serions alors forcés d'intervenir dans des conditions encore plus dégradées, comme nous l'avons fait contre les talibans ou contre l'État islamique. En somme, l'action militaire n'empêche pas la défaite ; la victoire demeure entre les mains des responsables politiques locaux. Rien, cependant, ne permet de dire quand de telles solutions pourront être trouvées. La France doit donc s'attendre à ce que son intervention dans la région dure- nous devons nous y préparer. Dans ces conditions, il convient de rendre notre effort soutenable. Il faudra continuer à chercher des soutiens concrets à l'action que nous menons, pour que nous ne soyons pas seuls à supporter les coûts de cette opération, qui sert les intérêts de tout le continent européen. Nous ne pouvons réduire notre effectif que dans la mesure où de nouveaux contingents européens prennent la relève. L'Europe doit prendre en considération cette dimension, soit par une mutualisation des coûts, soit par une contribution accrue à l'aide au développement des pays du Sahel. En effet, convenons-en ensemble, lutter contre la misère reste aussi le grand défi à relever. La parole est

Mis à part les débats budgétaires, n'autorisant aucune discussion stratégique, son rôle est réduit à néant. L'esprit de l'article 35 de notre Constitution s'est évanoui depuis bien longtemps ! Aussi, je me félicite de l'organisation de ce débat à la demande de notre commission, même si celui-ci n'engage nullement le Gouvernement. Il y a pourtant beaucoup à dire et à proposer ! Sept ans après le début de l'opération Barkhane, le bilan de l'engagement français nous laisse perplexes. Voilà un an, lors du sommet de Pau, le Président de la République annonçait une montée en puissance de l'opération, notamment par l'envoi d'un renfort de 600 hommes. Le coût financier de l'opération, lui aussi, s'est accru : de 520 millions d'euros en 2014 à environ 1 milliard d'euros en 2020. Pour quels résultats ? Certes, l'opération Barkhane engendre des succès tactiques, comme les opérations Bourrasque et Éclipse. succès nous rapprochent-ils des objectifs de la France et de ses partenaires ? Les armées locales sont-elles en capacité de circonscrire la menace terroriste ? Les États du Sahel ont-ils rétabli leur autorité et engagé un processus de réconciliation ? Si tels sont nos objectifs, nous en sommes encore loin ... En effet, il est clair que la neutralisation d'individus de haut rang ne fera pas disparaître le terrorisme sur le long terme. L'hybridation des groupes armés avec le tissu local et la montée des conflits communautaires sont nourries par des tensions systémiques, au premier rang desquelles, le changement climatique. La désertification, les sécheresses, qui déciment les cheptels et assèchent les points d'eau, touchent durement les éleveurs et les populations. L'insécurité alimentaire s'ajoute aux violences quotidiennes et permet aux groupes terroristes de proliférer. Face à ce bilan, les insuffisances de l'intervention militaire deviennent évidentes. Or ces insuffisances ont un coût humain, qu'il n'est plus possible de négliger. Je pense d'abord aux pertes parmi l'armée française. À ce jour, nous déplorons 55 morts français au Sahel depuis 2013 les derniers, le brigadier Loïc Risser et le sergent Yvonne Huynh, sont tombés au mois de janvier 2021, et je leur rends ici, ainsi qu'à leur famille, un hommage appuyé. Mais la population civile locale est la première victime de ces conflits. Les pertes civiles ne se comptent plus en centaines, mais en milliers de personnes, sans parler des millions de déplacés et de réfugiés. Dans un tel contexte, les circonstances de la frappe opérée le 3 janvier près de Bounti au Mali, qui aurait potentiellement touché des civils, doivent impérativement être éclairées. Cette transparence est nécessaire, car une intervention qui ne serait plus soutenue par la population locale perdrait sa légitimité. Nous sommes aujourd'hui à la veille du sommet de N'Djamena, où se réuniront de nouveau le Président de la République et ses homologues du Sahel pour un bilan d'étape. Ce bilan doit être un tournant, car l'enlisement, qui devait être à tout prix évité, semble déjà une réalité. À cet effet, il nous apparaît important de rappeler que la la solution militaire ne remplacera jamais la solution politique. Dans un contexte de démocratie fragilisée, voire absente depuis le coup d'État d'août 2020, il faut en priorité appuyer les transitions démocratiques et redonner un souffle à l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. À ce jour, malgré l'activisme affiché par l'Algérie à la fin de l'été, sa mise en oeuvre reste laborieuse. Les États et organisations médiateurs, avec, en tête, l'Algérie, la France et l'ONU, doivent donner ensemble une nouvelle impulsion à l'accord. ailleurs, le tabou des pourparlers avec certaines des organisations armées doit être débattu. Les négociations poursuivies par certaines personnalités maliennes avec ces groupes sont déjà une réalité et doivent être accompagnées par la France, lorsque les revendications politiques ou territoriales portées ne sont pas incompatibles avec nos exigences. À cette fin, la France doit soutenir l'évolution d'un cadre politique clair et légitime. Ensuite, si notre pays décide un désengagement progressif, celui-ci doit s'accompagner d'une participation européenne accrue et garantie par un renforcement du G5 Sahel. Malgré le lancement de la Takuba l'année dernière, la participation de nos partenaires européens reste trop limitée les contingents estoniens, tchèques et suédois intégrés à l'opération ne représentent pas une capacité supplémentaire décisive. Or, au vu de la responsabilité que portent nos voisins européens sur l'intervention au Sahel, une participation plus importante sur le volet développement serait entièrement justifiée.

La deuxième piste est celle qui demandera plus d'efforts, sans doute plus d'engagement à nos partenaires, à commencer par nos partenaires européens. Certes, Takuba est une avancée, mais celle-ci est insuffisante. La perspective la plus prometteuse

de mon point de vue- et, si je suis ici aux côtés de la ministre des armées, c'est que vous partagez ce constat -, on ne saurait traiter ces questions sans prendre en compte l'ensemble de l'architecture dans laquelle cette opération s'insère désormais, que nous avons patiemment bâtie au fil des années avec nos partenaires sahéliens, européens et internationaux. La création du G5 Sahel en 2014, la mise en place de sa force conjointe en 2017, celle de l'Alliance Sahel la même année, le lancement du Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, parfois appelé P3S, en 2019 et, enfin, la création de la Coalition pour le Sahel l'an dernier sont autant de jalons décisifs dans un double mouvement d'internationalisation de la lutte contre la menace terroriste au Sahel et de définition d'un cadre global et intégré pour apporter à cette crise complexe, non seulement les réponses du court terme, celles de l'action militaire et de la stabilisation, mais aussi les réponses du temps long, celles de la négociation politique et du développement. double mouvement montre que, depuis huit ans, les lignes ont considérablement bougé au Sahel, en dépit des polémiques sur un enlisement français dans cette région, polémiques qui, elles, n'avancent guère.

de pointer trois malentendus qui planent encore trop souvent sur les discussions que nous pouvons avoir sur le Sahel, dont, j'espère, nous saurons nous garder aujourd'hui- vous l'avez fait jusqu'à présent, j'ai pu le constater en vous écoutant. Le premier de ces malentendus tient à une forme d'amnésie

rappeler les raisons de notre engagement, d'abord dans le cadre de l'opération Serval, puis dans le cadre de l'opération Barkhane. Comme vous le savez, en 2012, le Mali se trouvait au bord de l'effondrement

puisqu'une alliance de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda occupait le nord du pays jusqu'à Tombouctou, où ces groupes avaient entrepris de soumettre la population locale à la charia et de détruire la charia et de détruire des mausolées classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Ils se préparaient à prendre d'assaut la capitale du Mali, Bamako. Cet effondrement aurait été une véritable catastrophe, non seulement pour la population malienne, qui aurait été condamnée à vivre sous la loi d'un califat islamique implacable, mais également pour nous, en France et en Europe, puisque ce califat aurait pu servir de sanctuaire aux djihadistes un sanctuaire où attirer des combattants en provenance de l'étranger, un sanctuaire d'où il aurait été possible de projeter des attaques vers l'étranger. Je vous rappelle que, un an et demi plus tard, au Levant, d'autres djihadistes, toujours de la même obédience, proclamaient l'instauration d'un proto-État totalitaire, le pseudo-califat de Daech. Nous avons donc eu raison, chacun l'a souligné, de prendre cette menace très au sérieux et nous avons eu raison d'agir très vite en lançant l'opération Serval dès janvier 2013, à la demande

un coup d'arrêt à la progression des djihadistes vers le Sud et a permis de libérer les régions du Nord. Sur le plan politique, cette opération a aussi permis le retour d'un processus démocratique avec l'élection du Président de la République du Mali, laquelle s'est déroulée dans de bonnes conditions. Mais, parce qu'ils avaient été défaits au Mali, nos adversaires sont passés d'une stratégie d'implantation locale que je serais tenté d'appeler « stratégie d'occupation territoriale » à une stratégie de déstabilisation régionale. Si bien que la menace terroriste s'est étendue à l'ensemble du Sahel. C'est pourquoi, en août 2014, nous avons lancé l'opération Barkhane afin de nous donner les moyens de limiter leur liberté de mouvement en intervenant à l'échelle de la région tout entière

unies. Le deuxième malentendu tient, justement, à une forme de myopie qui pourrait conduire à voir le Sahel comme une affaire franco-française, pour ne pas dire une obsession française, comme on l'entendait naguère. Ce n'est pas le cas les 5 100 femmes et hommes de Barkhane ne sont pas seuls sur le terrain. La sécurité du Sahel, c'est évidemment d'abord l'affaire des États du Sahel, et notre stratégie a toujours consisté à appuyer la montée en puissance de leurs armées nationales et de la force conjointe- la ministre des armées y reviendra tout à l'heure -, parce que c'est le levier de leur future sécurité. De fait, nous n'avons pas vocation à rester là-bas pour l'éternité. Il faut donc faire en sorte que ces outils se construisent progressivement : c'est ce que nous faisons. Si nous ne sommes pas seuls, c'est aussi parce qu'il y a eu une prise de conscience européenne- sans doute tardive.

Ils le sont avec la force Takuba, qu'évoquera Mme la ministre des armées ; ils le sont en appuyant la force conjointe de manière significative pour financer les équipements ; ils le sont dans le cadre des missions de formation EUTM et EUCAP ; ils le sont aussi dans le cadre de la mobilisation dans le cadre de la mobilisation internationale autour de la mission de maintien de la paix des Nations unies, la Minusma. J'ajoute que, année

on pourrait déplorer qu'une certaine forme d'impatience tende parfois à fausser l'appréciation de notre engagement au Sahel, comme si nos récents succès militaires pouvaient à eux seuls suffire à assurer le retour de la paix. Or, on le sait bien, le règlement de cette crise sera obligatoirement politique. Soyons clairs entre nous : si le Sahel est depuis huit ans en proie un tel degré d'instabilité et de violence, c'est en raison des fragilités considérables auxquelles doit faire face cette région, lesquelles ne pourront se résorber qu'étape après étape. La clé du succès, c'est donc la mise en oeuvre d'une approche globale et intégrée de la crise. Tel est le sens de la Coalition pour le Sahel, dont l'architecture, telle qu'elle a été définie au sommet de Pau du mois de janvier de l'année dernière avec avec les pays du G5 Sahel, s'appuie sur quatre piliers prioritaires, mais indissociables : la lutte contre le terrorisme ; le renforcement des capacités des forces armées sahéliennes le soutien au déploiement de l'État, des administrations territoriales et des services de base et la reconquête par les États de leur propre territoire ; le développement. Cette coalition

qui vient de nous rejoindre -sont déterminés à agir ensemble autour des États du G5 Sahel pour la sécurité et l'avenir des populations de la région. C'est une structure conçue dans un souci de pragmatisme, d'agilité. C'est un multilatéralisme nouveau, une sorte de consensus en acte de la communauté internationale, comme l'on dit, sur cet enjeu. Si bien que, un an après le sommet de Pau, le secrétariat de cette coalition est en train de s'installer à Bruxelles, pour en

dans le cadre de la politique de stabilisation- c'est le troisième pilier -et de développement- c'est le quatrième pilier. S'agissant du troisième pilier- le redéploiement des États et de leurs services

qui travailleront à consolider le contrôle des territoires arrachés à l'influence des djihadistes pour rétablir la présence de l'État dans les territoires ainsi libérés- c'est le cas en ce moment même au centre du Mali, où nous menons cette expérimentation. des progrès dans le renforcement de la chaîne pénale et dans la lutte contre l'impunité, l'un des engagements que nous avons pris en commun à Pau. L'appui apporté aux autorités judiciaires dans le traitement des dossiers du terrorisme a permis, par exemple, en octobre dernier, la tenue du procès des auteurs des attentats de la Terrasse et du Radisson Blu à Bamako. Ces progrès dans la lutte contre l'impunité sont réels, mais ils sont encore insuffisants. nous poussons les pays du Sahel à assumer pleinement leurs responsabilités et à faire toute la lumière sur les allégations d'exactions lorsqu'elles se produisent. progrès, s'agissant toujours de ce troisième pilier, dans la mise en oeuvre du redéploiement dans les zones libérées des administrations et des services de base, comme l'éducation, la santé ou encore l'état civil.

déminer, en même temps construire des écoles ou des centres de santé, il faut faire en sorte que les lieux où s'exerce symboliquement et concrètement l'autorité de l'État soient réhabilités et il faut aussi immédiatement mettre en place un accès minimal à l'eau et à l'électricité. Sur ces projets d'urgence,

pour rendre des perspectives d'avenir aux populations, pour traiter en profondeur les fragilités et pour inscrire le retour à la stabilité dans la durée. C'est pour cette raison que nous avons contribué à créer, en 2017, avec

avec un effort de concentration sur les zones les plus sensibles et les plus fragiles. Nous sommes évidemment très impliqués dans l'Alliance Sahel, qui tiendra d'ailleurs son assemblée plénière

développement a octroyé 480 millions d'euros aux pays du G5 Sahel et décaissé 350 millions d'euros en un an pour accélérer la mise en oeuvre des projets qu'elle finance dans le secteur de l'eau, de la santé et de l'éducation,

Se battre pour l'éducation, c'est aussi se battre contre l'obscurantisme et faire en sorte que les filles et les garçons du Sahel aient plus tard la liberté de choisir leur avenir. C'est donc encore une manière de combattre la menace terroriste, de tous les combats en faveur de la stabilisation et du développement engagés par la France, les Européens et la communauté internationale au Sahel. Quand plus de 5 millions de personnes retrouvent un accès à des services d'approvisionnement en eau, quand 3 millions de personnes bénéficient d'une assistance alimentaire, quand on propose à des centaines de milliers de femmes une méthode de planning familial dans une région en proie à une croissance démographique exponentielle-

le sommet de Pau a été le sommet du sursaut militaire, le sommet de N'Djamena doit être le sommet du sursaut diplomatique, du sursaut politique et du sursaut du développement

et les pays riverains du golfe de Guinée afin d'enrayer l'extension de la menace terroriste vers leurs territoires. C'est fondamental. Cette prise de conscience a lieu : le Président du Ghana a pris l'initiative dite « d'Accra », qui vise à vise à conforter la relation particulière entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Ghana pour solidifier la sécurisation du nord de ces pays. Cette initiative doit déboucher sur un accord opérationnel avec les pays du Sahel directement concernés et permettre de renforcer la protection des frontières nord de ces pays. Ce somment doit pour renforcer la coopération des pays du Sahel avec l'Algérie et le Maroc et pour faire le lien avec la question libyenne. Ensuite, le sommet de N'Djamena doit être un sursaut politique.

d'une meilleure représentation des populations du Nord au sein des instances nationales, dans le respect de l'unité et de l'intégrité du Mali évidemment, d'une refonte de l'armée malienne pour y intégrer des combattants des mouvements armés du Nord et d'un effort considérable de développement de ce Maintenant, il faut passer aux actes, mais cette interpellation vaut pour ceux qui siègent au comité de suivi des accords d'Alger, en particulier les acteurs de la zone, singulièrement ceux du Mali je pense à la nécessité de réinstaller l'armée malienne reconstituée à Kidal ; je pense à la poursuite du processus de désarmement-démobilisation-réintégration des ex-combattants

Cet accord est fondamental aussi parce qu'il établit une distinction politique claire entre les groupes armés signataires et les groupes terroristes.

dont l'objectif déclaré est de mettre à bas l'État malien. On ne négocie pas avec des terroristes, on les combat ! Il est également essentiel que la transition civile au Mali soit menée à bien.

que les demandes de réformes de la population malienne soient entendues, notamment en matière de gouvernance, de lutte contre l'impunité et de refonte du cadre et d'engagement face aux défis sécuritaires. Nous allons également proposer que N'Djamena soit le moment du sursaut de la stabilisation et du développement, pour gagner encore en réactivité et en efficacité face aux défis du long terme. Cela passe par une prise de responsabilité des États du G5 Sahel, appuyée par une meilleure coordination de l'aide de leurs partenaires internationaux, car, aujourd'hui, je dois le dire, la coordination et, surtout, la territorialisation de l'aide ne sont pas satisfaisantes. Il faut donc ouvrir davantage d'écoles, recruter davantage d'enseignants, créer et faire vivre davantage de dispensaires. Ces pistes concrètes seront au centre de nos échanges. Nous voulons aussi tirer profit du sommet de N'Djamena pour confirmer la relance que nous avons initiée du projet de grande muraille verte.

d'autres pays très actifs dans la zone tels que l'Allemagne et l'Espagne, au titre de sa présidence de l'Alliance Sahel, ainsi que nos partenaires britanniques, américains et canadiens au sein de Barkhane, l'Algérie, le Maroc, l'ensemble des Européens engagés dans la Takuba. petite communauté internationale qui se réunit à N'Djamena pour continuer à la fois la lutte contre le terrorisme et permettre de tracer les chemins de la paix pour l'ensemble des populations du Sahel, meurtries depuis maintenant de

mesdames, messieurs les présidents de commission et de groupe, mesdames, messieurs les sénateurs, en introduction de mon propos, je souhaite naturellement m'associer à l'hommage que vous avez tous rendu à nos militaires et avoir une pensée particulière pour la famille de Jean-Marie Bockel.

le Mali a fait appel à la France pour stopper des colonnes de djihadistes qui fonçaient sur Bamako. Nous avons répondu à cet appel, car c'est ainsi que nous nous comportons avec nos partenaires et c'est ainsi que nous souhaiterions que nos partenaires se comportent si nous étions un jour agressés. Nous avons répondu à cet appel pour protéger le Mali et sa population, mais aussi pour protéger les États sahéliens des groupes terroristes qui veulent les détruire et les soumettre pour imposer leur loi, terroriser et tuer tous ceux qui s'opposent à eux. Nous avons aussi répondu à cet appel du Mali, parce que, comme le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a rappelé, nous ne voulons pas que le Sahel devienne un sanctuaire terroriste, nous ne voulons pas qu'il leur permette de préparer des attentats dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, voire en Europe. Depuis huit ans, les forces armées françaises se sont sans cesse adaptées- certains ont dit « ajustées » et sera encore amenée à évoluer. Je voudrais maintenant revenir avec vous sur l'évolution de la stratégie de la France au Sahel que le Président de la République a opérée il y a un an au moment du sommet de Pau. Souvenez-vous, il y a un an, les forces armées sahéliennes étaient débordées de toutes parts, pour ainsi dire au bord de la rupture. En l'espace de deux mois seulement, le Niger avait enterré 160 de ses soldats, après les attaques d'Inates et de Chinagodrar, et le Mali 53 militaires et civils après l'attaque de la garnison à Indelimane. Il y a un an, on observait la montée du discours antifrançais, qui n'était pas clairement démenti, souvenez-vous-en, par certaines autorités des pays du G5 Sahel. Il y a un an, on observait aussi que la mobilisation des pays sahéliens n'était pas forcément à la hauteur des enjeux. Au milieu, il y avait un véritable boulevard pour Daech et Al-Qaïda au Sahel, qui multipliaient leurs actions et se renforçaient chaque jour davantage. Le Président de la République a donc convoqué un sommet avec l'ensemble de nos alliés et de nos partenaires pour revoir notre stratégie commune et pour s'assurer que la présence des armées françaises au Sahel était bien voulue et non pas subie. De ce sommet, je crois pouvoir dire que nous sommes sortis plus forts et plus nombreux. C'était en effet un message fort de solidarité avec les pays sahéliens, un message de remobilisation régionale et internationale dans la lutte contre le terrorisme. La création de la Coalition pour le Sahel- le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a rappelé -nous a offert un cadre d'action reposant sur quatre piliers

c'est la lutte contre le terrorisme, en particulier contre l'État islamique dans le Grand Sahara, affilié à Daech dans la région des trois frontières, cette région qui se situe à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est pour intensifier cette lutte que le Président de la République a décidé il y a un an de renforcer les effectifs de Barkhane de 600 militaires supplémentaires. Le second pilier, c'est la montée en puissance des forces armées sahéliennes. Depuis un an, ce sont ces deux objectifs qui ont guidé notre action. Au bout d'un an, des résultats significatifs ont été obtenus : l'effort militaire sur la zone des trois frontières a porté ses fruits. Daech au Sahel est fortement entravé, même s'il conserve encore une capacité de régénération importante. Concrètement, en 2019, 300 membres des forces de sécurité- garde nationale, police, gendarmerie ou militaires -avaient été tués en six mois. Si, depuis un an, nous déplorons près de 100 policiers ou militaires tués par des groupes terroristes au gré d'actions d'opportunité dans la région du Liptako, qui est à cheval entre le Mali et le Niger, il convient de noter que, depuis janvier 2020, plus aucune attaque d'ampleur n'a été commise. Nous avons également réussi à affaiblir Al-Qaïda en neutralisant son numéro un dans la région ainsi qu'un certain nombre de ses cadres. Par ailleurs, la montée en puissance des armées sahéliennes se confirme : nous observons chaque jour des progrès et des résultats encourageants. Au début de cette année 2021, à partir du 2 janvier très exactement, jusqu'au 3 février, près de 2 000 militaires des forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes, ainsi que de la force conjointe du G5 Sahel, ont conduit, au côté de la force Barkhane, une opération de grande ampleur baptisée Éclipse, qui a pris donc le relais de l'opération Bourrasque. L'ennemi a été bousculé et surpris par la rapidité de l'intervention. Face à la puissance des unités engagées, les groupes terroristes se sont repliés et ont abandonné de nombreuses ressources : des motos, des pick-up, des équipements de communication, ainsi que d'importants matériels et produits permettant la fabrication d'engins explosifs improvisés qui peuvent être si meurtriers, comme nous le savons si bien. Contrairement à il y a un an, les forces armées locales sont désormais capables de résister et de répliquer. Elles ne sont plus démunies face à la violence des attaques terroristes, même si, bien sûr, elles ont encore besoin d'être accompagnées. Cela est possible grâce à Barkhane, bien sûr, mais aussi et surtout grâce à un engagement international et européen qui s'est confirmé et renforcé. Je pense en premier lieu tout particulièrement aux Européens, aux Européens, dont l'engagement en faveur de la formation des forces armées locales est essentiel au travers de la mission de l'Union européenne EUTM Mali. Quand je dis qu'il y a des Européens au Sahel, on me pose à peu près systématiquement la question : « Mais où sont les Allemands ? je peux vous dire qu'ils sont là ! Ce sont même les deuxièmes contributeurs, derrière la France, à la mission de formation des forces armées maliennes de l'Union européenne. Partenaire européen de premier plan, l'Allemagne fournit 800 soldats au travers de ses déploiements au sein de la Minusma et de l'EUTM et elle devrait en fournir 450 de plus à la fin de l'année 2021 ou au début de Il y a aussi des Européens au sein même de Barkhane : des Espagnols, des Britanniques, des Estoniens, qui nous appuient par des moyens et des renseignements précieux. Un détachement danois a en outre renforcé Barkhane pendant toute l'année 2020. l'année 2020. Naturellement, le soutien américain contribue lui aussi au succès de nos opérations. Plus récemment, nous avons mis sur pied une force composée de forces spéciales européennes, entièrement consacrée à l'entraînement et à l'accompagnement au combat des forces armées maliennes : c'est la force Takuba. Cette force est aujourd'hui composée d'un groupe de forces spéciales franco-estonien, d'un groupe franco-tchèque et d'un détachement suédois composé de 150 militaires, qui, au moment où je vous parle, est en train de se déployer. fournissent des capacités aéromobiles essentielles et une unité de réaction rapide. D'autres nations sont prêtes, elles aussi, à s'engager.

en engageant un contingent dans Takuba, ces pays acceptent d'aller au combat. Ils acceptent le contact direct avec l'ennemi. Ce sont des alliés qui ont compris que la stabilité du Sahel était clé pour la sécurité européenne. Ils sont prêts à se battre auprès de nous pour lutter contre le terrorisme. Leurs contributions- vous en conviendrez -sont tout sauf insignifiantes. Si des Européens s'engagent aujourd'hui à nos côtés, c'est parce qu'ils croient au sens de cet engagement. C'est aussi parce que la France y est et que l'organisation et le savoir-faire de nos armées facilitent la présence d'armées moins puissantes. Je l'ai dit et je le répète : Barkhane n'est pas éternelle. Mais à court terme nous allons rester, ce qui n'exclut pas que les modalités de notre intervention évoluent- s'ajustent, diraient certains -, bien au contraire. Les pays sahéliens souhaitent que nous continuions à les aider ; les résultats obtenus nous permettent d'accentuer la stratégie d'accompagnement des forces locales avec nos partenaires et avec nos alliés sur le terrain. le contre-terrorisme au Sahel est et reste une priorité, contre Daech et contre Al-Qaïda. Comme le rappelait Bernard Emié, directeur général de la sécurité extérieure, il y a quelques jours, à la sortie du comité exécutif ministériel que nous avons consacré au contre-terrorisme, le risque d'expansion du djihadisme vers le golfe de Guinée et l'Afrique de l'Ouest est réel. Certains d'entre vous l'ont souligné. Le projet politique qu'il y a derrière est clair : faire de la région la base arrière du djihadisme. Notre enjeu est donc de réussir à transformer les gains et les victoires tactiques en progrès politiques, économiques et sociaux, tout en adaptant sans cesse notre engagement, de façon collective et concertée. Ce sera tout l'objet du sommet de N'Djamena qui se déroulera la semaine prochaine. Nous allons

avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

Il existe au Sahel un vrai risque de contagion vers le golfe de Guinée, qu'il faut absolument contenir. La menace étant mondiale, notre réponse doit également être d'ampleur internationale. Dans cette guerre contre le terrorisme, nous ne sommes pas seuls. Avec nos partenaires européens, pas assez nombreux, hélas ! et des alliés sahéliens, nous luttons contre l'ennemi commun. À mon sens, l'exemple de la force Takuba, pilotée avec certains partenaires européens, a permis de montrer la puissance de la coopération entre les nations pour éliminer cette menace qui nous est commune. En partageant nos connaissances avec les forces militaires locales, nous allons dans le sens d'une sécurisation pérenne sur le long terme. Cet entraînement permet désormais aux forces sahéliennes, qui constituent le deuxième pilier du sommet de Pau, de monter en puissance, et les résultats sont encourageants. L'opération Éclipse,

dont 1 500 de la force Barkhane, auxquels s'ajoutent 1 900 soldats sahéliens- 900 Burkinabés, 850 Maliens et 150 Nigériens. Ces chiffres témoignent de l'envergure de cette opération conjointe menée avec nos forces partenaires. Vous l'avez dit en commission des affaires étrangères il y a quelques jours et vous l'avez rappelé à l'instant, madame la ministre : « Jamais nous n'avons vu les forces maliennes et nigériennes mener le combat comme cela a été le cas pendant les opérations de fin 2020 et notamment à travers l'opération Éclipse. Éclipse. » Pourriez-vous revenir sur le bilan opérationnel d'Éclipse et nous expliquer en quoi il confirme un changement profond ? Avec ce retour d'expérience, quels enseignements pouvons-nous d'ores et déjà tirer quant aux étapes à franchir pour que les armées sahéliennes puissent intervenir avec de plus en plus d'autonomie, puisque Barkhane ne sera pas éternelle ? La parole

Il y a eu, à la fin de l'année 2020, l'opération Bourrasque. Il y a eu, à compter du 2 janvier de cette année, l'opération Éclipse, dont vous avez rappelé l'ampleur : elle a mobilisé 3 400 militaires, dont 1 500 Français et près de 2 000 soldats partenaires. À ce titre, je souligne le retour des militaires burkinabés, qui n'étaient pas intervenus dans le cadre de l'opération Bourrasque. Le résultat s'est révélé probant : neutralisation de nombreux terroristes djihadistes, saisine et destruction d'un volume important de ressources logistiques. Quelles conclusions faut-il en tirer ? Cette stratégie, que je qualifierais de partenariat de combat,

Takuba. Je le répète, les Sahéliens se renforcent et contestent le terrain aux groupes armés terroristes. Nous en avons encore eu un exemple à la fin du mois de janvier dernier, avec les attaques menées contre Boulikessi et Hombori : les forces armées sahéliennes ont

de professionnaliser ces armées : c'est ce à quoi nous allons nous employer à leurs côtés.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat a reçu en audition M. Aguila Saleh, président du parlement de Tobrouk. M. Saleh nous a présenté la situation de son pays et les relations ambiguës que le gouvernement de Tripoli, dont il ne reconnaît pas la légitimité, entretient avec la Turquie. Il a notamment évoqué le détournement du produit de la vente du pétrole libyen au profit du financement de milices ou de mercenaires qui sévissent sur ce territoire. Un de ses objectifs, bien légitime, est de mettre un terme, après avoir démocratiquement repris le contrôle du pays, aux actions de ces milices ou de ces mercenaires, installés avec la complicité de la Turquie et avec la connivence du gouvernement de Tripoli. Dans le même temps, plus au sud, nos soldats se battent contre un ennemi diffus, sur un territoire immense. Ils sont confrontés à des attentats et à des embuscades lâches et meurtriers.

ce rappel à l'intention de ceux qui, constamment, comparent aveuglément notre déficit public à celui de nos voisins. Pour ce qui concerne le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ne craignez-vous pas, monsieur le ministre, que ces milices ou ces mercenaires, une fois empêchés d'intervenir en Libye, ne viennent renforcer d'une manière ou d'une autre les groupes armés terroristes au Sahel, mettant de fait

au Sahel. Nous arrivons au bout de notre modèle d'action fondé avant tout sur le militaire, malgré des concepts comme les « 3D » ou le continuum sécurité-développement. Se pose dès lors la question de nos perspectives en matière de développement et de diplomatie. Le 10 décembre dernier, le bureau du conseiller spécial pour l'Afrique de l'ONU, ses représentations permanentes de l'Afrique du Sud et du Nigéria ainsi que l'Union africaine ont présenté une nouvelle note sur les flux financiers illégaux en Afrique. Ce document, s'appuyant sur la feuille de route de Lusaka, prise sur l'initiative de l'Union africaine en 2016, dresse un tableau essentiel de la situation et des objectifs à atteindre. Ainsi, les flux financiers illégaux participent chaque année à la fuite de 88,6 milliards de dollars du continent. Cette somme représente presque autant que les rentrées annuelles combinées de l'APD et des investissements étrangers en Afrique ; ce sont autant de milliards d'euros qui maintiennent les États dans une situation de sous-développement et aggravent la pauvreté, facilitant d'autant le recrutement des groupes armés terroristes et créant des conflits entre les communautés. Parmi les recommandations de ce document, on retrouve des éléments centraux, comme la suppression des paradis fiscaux, qui permettent un accès rapide aux richesses illégalement acquises, mais aussi un renforcement des dispositifs de restriction de circulation des armes. De plus, la question de l'opérationnalisation du fonds spécial de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme est posée. Enfin, cette feuille de route fait de la lutte contre la corruption, du renforcement institutionnel des États et du renouvellement des élites politiques une priorité.

Madame la sénatrice, la question que vous abordez n'est pas spécifique au Sahel, même si le Sahel, comme les autres régions d'Afrique, est concerné par ce phénomène gravissime que constituent les flux financiers illicites. Vous avez raison de citer le rapport de la Cnuced, qui met l'accent sur ces dérives considérables et ces trafics inacceptables.

et ancien collègue Jean-Marie Bockel, ainsi que pour sa famille. Je remercie M. le président Cambon d'avoir rappelé que le lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel aurait dû fêter ses trente ans aujourd'hui. Nous souhaitons rendre hommage aux 55 militaires français tombés au combat et aux centaines de victimes que l'on déplore dans les rangs de nos alliés du G5 Sahel. Eux aussi paient un lourd tribut pour le rétablissement de la paix dans leur région.

Ils reconnaissent la prouesse militaire de l'armée française, que je veux saluer ici, faisant énormément avec si peu pour un si vaste territoire. Lors de ma première visite à Ouagadougou, il y a quatre ans,

notamment entretenu avec M. Roch Kaboré, Président du Faso. Il considère que le combat mené par les États de la région vise à contenir la menace, l'extension du phénomène en direction des pays côtiers se faisant sentir. la carte « conseils aux voyageurs », ces pays- Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana, Togo, etc. -affichent actuellement la même couleur que le Burkina Faso il y a quatre ans. La France envisage-t-elle des initiatives diplomatiques pour aider les pays côtiers à anticiper la menace terroriste qui les vise directement et pour accroître leur coopération militaire avec les pays du G5 Sahel ? Pour décrire la situation de son pays, le président de l'Assemblée nationale du Burkina, M. Alassane Bala Sakandé, a employé l'image d'une digue. Pour que la digue tienne, il faut que l'économie tienne. À Bamako, nos entrepreneurs me faisaient remarquer qu'il est moins cher et trois fois moins long de transporter un conteneur de France à Dakar que de Dakar à Bamako. La France compte-t-elle favoriser la création de corridors commerciaux depuis ces pays enclavés vers la mer, en relançant par exemple le Dakar-Bamako ferroviaire, à l'arrêt depuis 2018 ? je vous remercie

Il me semble important qu'une fois l'an la Haute Assemblée puisse mener un tel débat avec les deux ministres concernés, lorsque nos militaires sont engagés en opération extérieure. Fallait-il intervenir ? À l'évidence, oui ! Notre pays ne pouvait détourner honteusement le regard devant cette impérieuse nécessité. La France peut-elle rester éternellement ? Assurément, non ! En effet, chacun s'accorde à dire que ce conflit, comme bien d'autres avant lui, ne se gagnera pas militairement, mais politiquement. Or l'histoire nous enseigne que, si une intervention militaire ne s'accompagne pas d'un regard sur l'évolution démocratique, puis économique, sociale et enfin éducative, elle ne peut avoir d'effet durable. ceux qui nous ont applaudis à notre arrivée manifesteront quelques années plus tard pour nous demander de partir. S'agissant de l'évolution démocratique, nous savons que le népotisme habituel était resté, malheureusement, présent. Notre assistance continue ne mériterait-elle pas aussi d'être considérée en fonction des réels soutiens apportés, ou non, par nos partenaires occidentaux ? Sans eux, la France, seule, a-t-elle réellement les moyens de son ambition ?

Cet aspect géopolitique devient majeur. Dans ce nouveau cadre, pensez-vous que les États-Unis, qui nous aident militairement aujourd'hui, puissent renforcer leur soutien et accompagner la France, mais aussi l'Europe, pour éviter que le continent africain ne devienne étroitement dépendant de l'influence russo-chinoise grandissante ? La parole est à M. le ministre.

représentera une véritable coopération de pays volontairement et profondément associés à notre effort,

Voulez-vous l'associer, pour la mettre au défi de prendre ses responsabilités, au-delà du simple discours idéologique ? Je vous pose la même question s'agissant de la Russie, curieusement passionnée par la RCA,

le terrain. Ensuite, il faut des moyens. Les contingents qui viennent des forces spéciales européennes doivent être accompagnés d'équipements significatifs ; j'ai évoqué le contingent suédois, qui arrive avec des hélicoptères, ou le contingent italien, qui apporte des moyens d'évacuation sanitaire. C'est indispensable pour l'autonomie de la force Takuba.

Nous avons assisté en 2020 à de grands bouleversements. La pandémie a causé de nombreux morts, elle a aussi entraîné de graves conséquences économiques : la France a vu son PIB reculer de 8 % l'année dernière. Les conséquences de la crise continueront de se faire sentir dans les prochaines années. Parallèlement, la situation internationale connaît toujours un climat de tension dans lequel les menaces se multiplient et changent de formes. Plusieurs États se sont montrés agressifs à l'égard de l'Europe et de la France, et nous avons aussi constaté le développement d'organisations non étatiques hostiles. Le monde de demain ne sera pas moins dangereux que celui d'hier. Face à cela, de nombreux pays, dont la France, ont choisi d'augmenter significativement leur budget militaire. Boris Johnson a également annoncé que son pays allait investir 2,2 % de son PIB dans sa défense pour les quatre années à venir. Le Parlement a soutenu l'adoption de la loi de programmation militaire portée par le Gouvernement afin de redonner à nos militaires les moyens d'assurer la sécurité de la France dans de bonnes conditions. Cette loi doit cependant faire l'objet d'actualisations, dont une doit être mise en oeuvre avant la fin de l'année 2021, comme le précise son article 7. L'opération Barkhane nécessite un budget de plusieurs centaines de millions d'euros qu'il faudra maintenir, malgré la dégradation de la situation économique de la France. La France ne peut cependant pas assumer seule la défense de l'Europe hors de nos frontières. Les pays membres de l'Union européenne semblent encore bien loin d'avoir pris conscience de la nécessité de parvenir à une autonomie stratégique commune, même si certains d'entre eux participent à l'effort. L'unanimité sur le sujet paraît inatteignable. Sur Barkhane comme sur les autres aspects de la défense commune, plus encore à l'heure du départ des Britanniques, comment le Gouvernement et le Président de la République comptent-ils faire progresser la défense de l'Europe à l'avenir ?

des menaces auxquelles nous étions confrontés. Celles-ci n'ont pas faibli. J'aurai l'occasion, si le président de votre commission m'y invite, de venir présenter devant vous les travaux d'actualisation que nous avons conduits récemment et qui viennent d'être publiés. La réponse à ces menaces est, bien sûr, la préparation de nos armées, sous-tendue par cette loi de programmation militaire, mais aussi la construction de partenariats. À la veille de la présidence française de l'Union européenne, il est certain que nous devons continuer à encourager les Européens à prendre conscience

d'une nouvelle administration américaine et l'influence que cela peut avoir sur la manière dont nos partenaires européens vont répondre à ce besoin d'une Europe de la défense plus structurée et plus puissante. plus puissante. Pendant les quelques mois qui nous restent avant le début de la présidence française, nous entendons continuer à promouvoir les notions d'autonomie stratégique et de souveraineté européenne, car l'expérience récente nous a appris que, même si notre partenaire américain se réengageait dans un cadre multilatéral, il était important que nous apportions, en tant qu'Européens, la démonstration de notre engagement pour défendre notre sécurité et celle de nos concitoyens.

Un rééquilibrage des moyens financiers en faveur de l'aide publique au développement est indispensable. Nous l'avons déjà constaté, entre 800 millions et 1 milliard d'euros sont dépensés chaque année pour l'opération militaire Barkhane ; à titre de comparaison, seuls 400 millions d'euros d'aide au développement ont été dépensés entre 2013 et 2017 pour le Mali. De surcroît, nous nous interrogeons sur les modalités de mise en oeuvre des projets. Quel est réellement l'impact de cette aide sur les populations auxquelles elle est destinée ? Les efforts faits pour améliorer la traçabilité des flux financiers, notamment dans le cadre de l'Alliance Sahel, initiée avec l'Allemagne, aboutissent-ils à de réels changements ? Enfin, si les projets de développement restent ponctuels et peu suivis et servent en premier lieu à assurer aux forces armées françaises le soutien des populations, leur mise en oeuvre ne sera qu'un paravent de la situation socio-économique très dégradée dans la région. Nous soutenons que la mise en oeuvre de véritables programmes de développement au plus près des intérêts des populations est une priorité pour la sortie de crise. Ce point est fondamental. Plus que le djihad, c'est la situation économique et sociale qui fournit le terreau permettant aux organisations terroristes de perdurer, voire de se renforcer. J'ai notamment à l'esprit le pastoralisme, absolument essentiel pour l'économie sahélienne, qui est aujourd'hui menacé par l'avancée du désert et la raréfaction de l'eau, mais également les coopératives, souvent organisées par les femmes, qu'il faut soutenir. Vous l'avez compris, seul un effort considérable et ciblé de soutien aux populations locales permettra de créer les conditions nécessaires à la diminution des tensions communautaires.

débouchés existent, notamment l'opération grande muraille verte, lancée au Sahel en 2007 et qui patine, faute de moyens suffisants. Ce projet ambitieux vise à stopper la progression du Sahara en plantant des forêts à sa lisière.

Depuis huit ans, l'armée française opère sur un territoire en proie à des trafics qui s'intensifient en raison de la porosité des frontières. Nos soldats, auxquels nous témoignons un soutien indéfectible, opèrent sous la menace constante d'embuscades ou d'engins explosifs improvisés. La France s'inscrit, avec les pays membres du G5 Sahel, dans une coalition de régimes politiques et militaires avec pour objectif de lutter contre les groupes armés terroristes. Consciente que l'avenir de cette région passe par l'implication des pays de la zone, la France développe au maximum les différents aspects de la coopération interétatiques. la montée en puissance des forces armées nationales est contrastée, selon les derniers rapports de la Minusma et d'Acled, qui rappellent que, en comptant les groupes d'autodéfense, celles-ci sont responsables de plus de 70 % des décès au Mali. Face à la multiplication des protagonistes, l'enjeu, pour les gouvernements de la région, est d'encadrer ces milices, parfois proches des États. Enfin, la position française est d'autant plus compliquée que la population malienne commence à se retourner contre notre présence. Le 3 janvier 2021, nos forces ont été accusées de bavure à côté de Bounti. Cette même accusation a été relayée sur les réseaux pro-russes et pro-turcs. À l'heure où 50 % des Français sont encore favorables à l'opération Barkhane et face à la potentielle dégradation de l'image de la France malgré les efforts consentis, avant tout sur le plan humain, mais aussi financièrement, il est urgent d'établir un agenda politique. Ainsi, quelles vont être les mesures prises pour créer les conditions de la stabilité dans cette région et les indispensables évolutions politiques, tout particulièrement au Mali L'Union européenne envisage-t-elle une stratégie plus intensive d'aide au développement, pour faire reculer la pauvreté et le ressentiment, ferments du recrutement des mouvements islamistes ? Monsieur le sénateur, vous avez quasiment repris l'ensemble des sujets qui ont été évoqués au cours de ce débat. Il m'est difficile de sélectionner tel ou tel aspect. Je connais bien la région.

Rapidement, dès les premières années de son déploiement, l'opération Barkhane a mobilisé sur place plus de 3 000 soldats, puis près de 4 500 à compter de 2018. À la suite du sommet de Pau, 600 soldats supplémentaires ont rejoint leurs camarades de combat. Cette mission est légitime et utile, disons-le sans nuance.

la mission de formation de l'Union européenne aide à la reconstruction de l'armée malienne et les pays de la région ont formé utilement la coalition du G5 Sahel. Certes, la force Takuba permet l'implication sur le terrain d'armées nationales européennes qui ne sont d'ailleurs pas forcément les plus dotées, notamment celles de l'Estonie, de la République tchèque et de la Suède.

Je le dis sans oublier qu'il y a eu des morts américains, mais aussi néerlandais, suisses et asiatiques dans le cadre de la mission onusienne. Nous saluons leur mémoire. Ces tristes contributions sont cependant sans commune mesure avec nos pertes et celles des Sahéliens. Je crains que les renforts italiens et grecs annoncés récemment, s'ils sont très bienvenus, ne suffisent pas à rééquilibrer le fardeau. Ma question est double. Premièrement, comment pouvons-nous nous contenter encore, s'agissant de Takuba, du simple soutien

Pour le dire autrement, exigerez-vous de nos partenaires européens un doublement, un décuplement ou une augmentation à la marge de leur aide actuelle ?

Cependant, il est vrai aussi que, si nous partions demain, les pays du G5 Sahel rencontreraient d'immenses difficultés à assurer par eux-mêmes l'intégrité de leurs territoires et la sécurité de leurs populations. Les groupuscules proches d'Al-Qaïda et de Daech auraient alors les mains libres. Sur le long terme, c'est la sécurité de nos concitoyens sur le sol français qui serait menacée par des attentats perpétrés depuis ce nouvel épicentre de l'islamisme radical. Que nous manque-t-il, alors, pour assurer le succès définitif de l'opération Barkhane, qui permettrait le retrait de nos troupes ? Pour faire face à la menace terroriste, nos alliés africains ne peuvent faire l'économie des défis institutionnels, économiques, éducatifs et sanitaires qui s'imposent à eux. Nos victoires militaires doivent aller de pair avec le déploiement de services publics stables, l'avènement d'une économie plus saine, la formation de forces armées et de sécurité performantes, le développement d'entreprises et d'écoles. Cette vision est au coeur de l'approche « 3D », pour diplomatie, défense et développement. Aujourd'hui, force est de constater que le troisième « D », celui du développement, fait défaut. J'ai bien entendu vos propos, monsieur le ministre, mais les chiffres publiés par l'OCDE sont éloquents : les pays du Sahel sont fléchés comme prioritaires pour l'APD française, pourtant, aucun d'eux ne fait partie des douze premiers bénéficiaires de nos aides. D'autre part, comment expliquer que les cinq pays sahéliens ne perçoivent que 4,5 % du montant des aides françaises, alors que le Maroc en dispose à lui seul de 5 % ? Nous avons consacré d'importants moyens au volet militaire et peu, en proportion, à celui du développement. Il est nécessaire de mener une véritable stratégie d'aide aux pays du Sahel, corollaire essentiel à l'action de nos armées. Ces interventions pourraient, en outre, mobiliser plus efficacement nos partenaires européens, qui peinent parfois à nous apporter leur soutien sur le plan militaire. En clair, madame la ministre, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'en complément des actions militaires, le temps est venu de mettre en oeuvre un Barkhane du développement ?

Conway-Mouret. Je souhaite à mon tour rendre hommage à celles et ceux qui consacrent leur vie, parfois, malheureusement, jusqu'au sacrifice ultime, à notre protection. Deux ministres, deux questions ; la première s'adresse à Mme la ministre des armées. Nos militaires déployés dans l'opération Barkhane au Mali depuis plus de huit ans mènent une guerre asymétrique contre le terrorisme. Sur le terrain, ils vivent quotidiennement sous la menace d'engins explosifs improvisés, à chaque sortie de leur base, dans des véhicules blindés légers, les plus adaptés aux missions, mais qui sont vulnérables et vieillissants. Les kits de surprotection des VBL MkI vont bientôt être livrés, mais avons-nous une feuille de route pour lutter efficacement contre les IED ? N'est-il pas temps d'engager une réflexion sur le compromis nécessaire entre mobilité, discrétion et protection pour les VBAE, peut-être faut-il la mener avec notre partenaire belge ? Par ailleurs, compte tenu de la mutation de la forme des combats, ne devrions-nous pas nous reposer davantage sur le support aérien et procéder ainsi à un rééquilibrage de nos forces pour continuer à exercer une pression maximale sur nos ennemis ? maximale sur nos ennemis ? Monsieur le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, vous avez rappelé, très justement, le consensus qui se dégage autour de l'idée que la résolution de la crise malienne passera surtout surtout par une approche globale liant défense, diplomatie et développement, qui permettra la reconstitution d'un État de droit. La population, qui ne voit guère les progrès que son pays devrait faire grâce aux centaines de millions d'euros que nous investissons dans de nombreux projets par le biais de l'aide publique au développement, continue de sombrer dans la pauvreté. Les bénéficiaires en sont les groupes armés, qui s'appuient sur une forme d'assise populaire pour renouveler leurs forces tombées au combat. Le véritable enjeu est donc bien de tarir la source de recrutement de ces groupes, qui attirent à eux, non pour des raisons idéologiques ou religieuses, une jeunesse sans espoir d'insertion économique et sociale, sans espoir d'avenir.

n'y reviendrai pas. Le démantèlement d'une partie des capacités d'IED a été réalisé. Nous ciblons les poseurs de ces engins et les réseaux.

depuis celui de Nouakchott, de ce que chaque pays consacre, en moyens humains et financiers, à la paix. Madame la ministre, depuis votre entretien avec votre homologue le secrétaire d'État américain, Lloyd Austin, Austin, avez-vous pu obtenir plus d'informations sur le niveau de participation des États-Unis dans la bande sahélo-saharienne en termes de drones, de renseignement et de transport logistique ? Sans ce soutien, nous savons que des opérations peuvent être compromises. À N'Djamena, une question de fond doit être clairement posée : point de vue, il est moins question d'agenda de retrait que de responsabilités. Nous ne gagnerons pas la paix sans déconstruire la propagande des djihadistes, qui étendent leur politique d'influence, de déstabilisation et de recrutement vers le golfe de Guinée, sans gagner la confiance des populations. Ce sommet doit être aussi un moment de franchise : l'excellence des diplomaties africaines n'ignore pas la présence de nombreuses influences étrangères. Il n'est pas inutile de rappeler que celles-ci n'ont ni les mêmes méthodes de résolution de crises ni la même appréhension des droits humains. Le très regrettable épisode dans le village de Bounti et les accusations proférées desservent la paix et favorisent les terroristes. Nos partenaires africains savent combien l'information est une bataille en soi. Monsieur le ministre, quel message la France portera-t-elle pour que chaque partie assume ses responsabilités, s'agissant notamment du respect des missions des soldats français ?

L'opération Barkhane au Mali joue un rôle déterminant dans la lutte contre le djihadisme et le terrorisme au Sahel, mais aussi pour notre sécurité, ici, en France et en Europe. En plus de pacifier la région du Sahel, Barkhane participe à la protection de notre démocratie et de la civilisation européenne. Je salue les hommes et les femmes qui engagent leur vie pour la France dans la lutte contre le terrorisme. Je soutiens nos forces armées et je rends hommage à nos morts. hommage à nos morts. À l'heure où la sécurité des Européens reste menacée par le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne et alors que la France est désormais la seule puissance militaire complète et indépendante au sein de l'Union européenne,

Par ailleurs, le Fonds européen de défense, qui se substitue au plan de développement industriel de défense, a vu sa dotation initiale divisée par deux : de 13 milliards, elle est passée à 7 milliards d'euros. Dans quelle mesure ce fonds assure-t-il un soutien à la France dans ces opérations ? Comment favoriser le dialogue entre États membres pour qu'ils soutiennent davantage encore l'effort militaire considérable consenti par la France contre le terrorisme islamiste au Sahel ? Sahel ? Enfin, la présidence française de l'Union européenne en 2022 devrait être l'occasion d'une prise de conscience en faveur de la défense de l'Europe et d'une participation accrue de tous aux opérations de paix. Comment préparez-vous d'ores et déjà cette échéance ?

pour lutter contre les groupes armés salafistes djihadistes, après avoir dû intervenir pour éviter la faillite des structures étatiques. De Serval à Barkhane, nos soldats sont l'honneur de la France et des acteurs de paix pour tous les pays de la zone ! La représentation nationale les soutient autant qu'elle en est fière. Reste que, au regard des moyens investis, ces explications et une évaluation de notre action sur place sont indispensables, tant pour nos compatriotes que pour les pays africains impliqués. Au fil des années, les critiques sont aisées ; mais dans quel état politique la zone serait-elle aujourd'hui, si la France n'avait pas répondu favorablement à la demande d'assistance et d'intervention du gouvernement malien ? présence ne saurait être considérée comme une occupation, alors que nos soldats protègent la population et forment les forces de sécurité locales pour permettre aux pays concernés de renforcer leurs structures étatiques face au terrorisme. L'un des objectifs du sommet de Pau était l'établissement d'un partenariat de combat pour intégrer les forces partenaires. Dans ce cadre, il a été convenu de concentrer les efforts, notamment pour améliorer la qualité de la formation des militaires des armées des pays du Sahel. Cet aspect de l'intervention est essentiel aussi parce qu'il conditionne un retrait progressif de nos troupes. Pourriez-vous dresser un bilan de la formation par les Français et de l'autonomisation des troupes maliennes ?

Heureusement, car tout doit être fait pour que ces appareils soient disponibles pour compléter l'intervention de nos forces au sol.

en permanence opérationnels ; nous surveillons cela comme le lait sur le feu.

Notre connaissance du théâtre est désormais assez précise, nos modes d'action se sont adaptés et les personnels se sont aguerris au contact d'une région et d'un ennemi rudes. Chacun d'entre nous ici a une pensée pour nos soldats tombés là-bas. Même si elles n'affrontent pas un État, nos troupes et leurs alliés africains font face à une adversité solide et organisée. Comme le commandant de l'opération Barkhane l'a rappelé, « l'ennemi a sa propre volonté : il aspire à un projet politique et dispose d'une stratégie pour le mettre en oeuvre Cet ennemi n'est pas unique, mais pluriel, protéiforme. Il est fait de différents groupes s'appuyant notamment sur les tensions communautaires, l'absence d'alternatives sociales et économiques et les difficultés des États de Il a su muter et s'ajuster à notre dispositif. Dans ce contexte, nous avons glissé d'une opération limitée à une véritable guerre asymétrique, qui s'installe dans la durée. L'opinion publique occidentale voit dans les modes d'action des ennemis une certaine lâcheté, quand d'autres y voient, au contraire, une efficacité redoutable, à moindre coût, pour atteindre leurs objectifs.

Merci, madame la ministre, pour ces précisions. Oui, la guerre asymétrique, le développement des technologies nivelantes et l'extension de la confrontation dans le champ informationnel mettent nos démocraties en difficulté dans leurs opérations. L'actualisation stratégique 2021 souligne bien « la généralisation du recours aux stratégies hybrides et multiformes Attirer au sol, sur leur terrain, des forces occidentales régulières est une vraie stratégie des groupes armés terroristes. Les armées françaises ont su faire évoluer leurs tactiques et leurs outils. Faisons, nous, évoluer notre doctrine d'information

dans le cadre d'une approbation d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et à reporter la caducité des plans d'occupation des sols (POS),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

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, en matière d'urbanisme, on pense souvent, à tort, que certaines mesures législatives relèvent d'ajustements techniques : l'urbanisme ne serait qu'affaire de technique ... Tel n'est pas le cas, comme nous le savons tous. À la vérité, comme les travaux en commission cette proposition de loi de mon collègue Rémy Pointereau soulève une question profondément politique, que je résumerai ainsi : souhaitons-nous une modernisation accompagnée, concertée, différenciée de nos politiques d'urbanisme local ou une transition à marche forcée, sanctionnée de recentralisation ? Rien ne reflète davantage la diversité de nos territoires que leurs documents d'urbanisme. renouvellement urbains, dite loi SRU, a instauré le plan local d'urbanisme (PLU), envisagé comme un nouveau document de référence pour les communes françaises. En réalité, la transition vers le PLU ne se fait que progressivement, pour des raisons que les élus locaux connaissent bien

il n'est pas facile de faire converger les visions de dizaines de communes. La transition vers le PLU avance, mais de nombreuses communes ont préféré rester régies par une carte communale ou, jusqu'à récemment, par un plan d'occupation des sols (POS). Il s'agit souvent de communes rurales de petite taille, qui ont fait ce choix par manque de moyens ou d'opportunités. Elles doivent être respectées et entendues.

au remplacement des cartes communales par les PLUi dans la loi, alors que celle-ci est aujourd'hui silencieuse. Nous savons, de la voix même des maires, que cette incertitude les place dans des situations délicates : d'abord, devoir conduire une seconde enquête publique ; ensuite, tomber sous le régime du règlement national sans l'avoir anticipé ; enfin, retarder l'entrée en vigueur des PLUi. Deuxièmement, cette proposition de loi tend à repousser de deux ans l'échéance de caducité des POS, pour la porter au 1 janvier 2023, afin que les dernières communes puissent faire aboutir leur nouveau PLUi. Malheureusement, l'ordre du jour parlementaire n'ayant pas permis d'examiner à temps ce texte, force est de constater que la caducité est bel et bien intervenue au début de l'année 2021.

en cohérence avec le projet de territoire ; le pragmatisme, ensuite, car j'estime qu'il n'était pas envisageable de remettre en vigueur les POS, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, de rétroactivité notamment- cela aurait engendré trop de contentieux. La commission a adopté quatre amendements traduisant ces principes. Tout d'abord, elle a ajusté la rédaction de l'article 1pour renforcer la procédure combinée introduite par l'auteur de la proposition de loi. L'abrogation de la carte communale et l'élaboration du PLUi pourront ainsi être menées de front avec des délibérations jointes et une enquête publique unique. C'est là davantage non seulement de sécurité, avec une abrogation explicite et articulée dans le temps, mais aussi de souplesse, avec une réduction des lourdeurs procédurales. à l'article 2, la commission a offert aux maires des communes frappées par la caducité des POS ce que nous avons appelé une « boîte à outils », afin d'en atténuer les conséquences les plus problématiques et d'améliorer le dialogue avec le préfet.

La première dérogation vise à restaurer le droit de préemption des communes dont le POS est caduc. Elles pourront ainsi continuer à constituer des réserves foncières pour mener leurs projets d'équipement collectif, de logement ou d'autres projets structurants. Les deux autres dérogations tendent à améliorer le dialogue entre le maire et le préfet et à favoriser le traitement au cas par cas des difficultés de terrain. Sous le régime du RNU, toute décision du maire relative aux autorisations d'urbanisme est soumise à l'avis conforme du préfet. Parfois, cela se traduit par des blocages

part, du recours à un sursis à statuer élargi, permettant d'attendre l'adoption du PLUi avant de statuer sur une demande : c'est une sorte de dérogation défensive. La commission a prévu, d'autre part, que les maires puissent solliciter du préfet l'usage de dérogations élargies

Madame la ministre, je conclurai mon propos en revenant sur les échanges que nous avons eus en commission. Certes, une partie des articulations que nous proposons auraient pu être apportées par un décret.

En outre, nombre des apports de la commission nécessitent de passer par la loi : restaurer le droit de préemption ; élargir le sursis à statuer ; modifier la procédure d'avis du préfet sur l'abrogation de la carte. En tant que législateurs,

C'est là tout l'intérêt de la navette parlementaire. Aussi, j'espère que le Gouvernement demandera l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, afin que la proposition de loi puisse poursuivre son chemin et apporter enfin aux élus locaux des solutions concrètes. que nous appelons de nos voeux vers des documents d'urbanisme plus concertés, plus respectueux de l'environnement, plus intégrés aux enjeux de logement et de développement économique, mérite un véritable accompagnement et des gages de confiance envers celles et ceux qui la conduisent au quotidien.

et aux POS, ces sujets essentiels pour l'urbanisme, tout particulièrement dans les zones rurales. Progressivement, les outils de l'urbanisme se sont en effet enrichis pour dépasser la seule utilisation du sol et devenir des éléments stratégiques de définition et de mise en oeuvre de projets de territoire ambitieux et équilibrés, intégrant à la fois les enjeux d'aménagement urbain, d'architecture et de paysage, de mixité sociale et de transition écologique.

Elles disposent aussi d'une palette d'outils, du plus simple au plus sophistiqué, en fonction de l'ambition du projet de territoire : nombre d'entre elles ont un PLU ou un PLUi

Avec l'augmentation des ambitions de leurs projets de territoire, les collectivités passent progressivement du RNU et des cartes communales au PLU ou au PLUi. Ainsi, depuis les années 2000, les POS ont progressivement laissé la place aux PLU. Il faut naturellement faciliter ces procédures et lever les incertitudes pour les collectivités,

Votre article 1 vise ainsi à préciser les règles de procédure applicables aux cartes communales. Mais, comme je l'ai indiqué devant la commission des affaires économiques le 27 janvier, quatre des cinq mesures que vous proposez sont déjà satisfaites. Je prendrai un seul exemple. Pour abroger une carte communale, l'autorité compétente est évidemment la collectivité qui détient la compétence d'urbanisme. Il ne paraît donc pas nécessaire de le préciser. Vous avez d'ailleurs, monsieur le rapporteur, proposé des amendements pour supprimer certaines des mesures déjà satisfaites. Je suis persuadée qu'il nous faut éviter de prendre des mesures redondantes. Je sais que cette conviction est très largement partagée, car l'inflation législative et normative complexifie inutilement la loi et, par conséquent, notre vivre-ensemble. Pour autant, les règles doivent être claires pour tous. À ce titre- c'est une ancienne enseignante qui vous le dit -, la pédagogie réside pour partie dans la répétition. C'est la raison pour laquelle je m'engage à envoyer une nouvelle instruction pour rappeler le cadre juridique existant à nos services déconcentrés, ainsi qu'aux collectivités. L'une des mesures que vous proposez répond, en revanche, à un réel vide juridique. Il existe en effet une période, de quelques jours à plusieurs mois, durant laquelle la carte communale est abrogée pour laisser place au PLU, alors même que ce dernier n'est pas encore en vigueur. Je me suis d'ores et déjà engagée en commission à régler ce problème, qui relève cependant d'un décret, et non de la loi. Ce projet de décret, monsieur le rapporteur, est déjà en cours de finalisation et pourra être pris assez rapidement. Soyez certain que je vous le ferai parvenir avant sa publication, afin que le Sénat

200 ont simplement lancé la procédure, sans passer les premières étapes, dans l'objectif de simplement prolonger leur POS. Vous avez donc fait le choix, monsieur le rapporteur, de remplacer la prolongation des POS par des mesures visant à empêcher que les projets se retrouvent bloqués dans les territoires. Je partage cette approche. Avant de décider de ne pas repousser la durée de validité des POS, je me suis évidemment assurée que cela n'aurait pas d'impact négatif sur les projets. Là encore, le droit en vigueur le garantit et permet d'opérer la transition en douceur. Le RNU n'empêche pas les projets dans les zones déjà urbanisées et, au cas par cas, hors des zones déjà urbanisées. ailleurs, les porteurs de projet ont également pu demander des certificats d'urbanisme permettant de conserver les règles du POS pendant dix-huit mois de plus. Vous avez souhaité compléter ce dispositif par deux mesures pour les communes qui seraient revenues au RNU, auxquelles je ne souscris pas. Tout d'abord,

permettre au préfet de déroger au RNU pour tout projet d'intérêt communal afin d'éviter de bloquer certains projets me pose également problème à plusieurs titres. cela est contraire au message porté par le Gouvernement au sujet de la lutte contre l'étalement urbain, dont nous mesurons tous les effets écologiques mais aussi économiques et sociaux dans nos territoires. cela pourrait être vu comme une recentralisation : le RNU permet à la commune de délibérer pour mobiliser des dérogations lorsque l'intérêt général est dûment justifié.

C'est en effet un outil stratégique pour récupérer les terrains nécessaires, au fur et à mesure de leur vente, en vue de réaliser des opérations d'aménagement. Compte tenu de son impact sur le droit de propriété, il convient de bien l'encadrer, notamment par rapport aux documents d'urbanisme en cours d'élaboration, et pas uniquement sur la base de l'ancien POS, ainsi que vous le proposez dans cette proposition

d'abord, nous rappellerons, d'ici au mois de mars, le cadre applicable à l'abrogation des cartes communales pour éviter toute difficulté de procédure. nous allons supprimer le vide juridique qui existe entre l'abrogation d'une carte communale et l'entrée en vigueur du PLU par un décret. du PLU par un décret. Nous avons déjà lancé la consultation des collectivités afin qu'elles nous fassent remonter les difficultés concrètes liées à l'abrogation des POS. nous mettons en place un groupe de travail avec les élus pour élargir le droit de préemption urbain pour les communes revenues au RNU. Je vous propose bien sûr, cher Rémy Pointereau, cher Jean-Baptiste Blanc,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la maîtrise de l'urbanisme par les communes constitue l'un des principaux acquis des lois de décentralisation. Elles contribuent ainsi à l'aménagement du territoire, dont la compétence doit être partagée entre les collectivités locales et l'État, garant de la cohésion des territoires et d'une vision d'ensemble. Les communes et les intercommunalités ont dû s'adapter à un droit de l'urbanisme marqué par une certaine instabilité pathologique le rendant particulièrement complexe à appréhender, ce qui suppose de recourir à davantage d'expertise. Dès lors, l'ingénierie territoriale conditionne l'exercice même de leur libre administration. Le transfert automatique de la compétence en matière d'urbanisme vers les intercommunalités, sauf minorité de blocage, prévu par la loi ALUR, combiné aux réformes territoriales successives à peine digérées, n'est pas aisé De plus, le paramètre financier n'est pas négligeable : les communes et EPCI font état d'importants points de blocage, au premier rang desquels le coût significatif de l'élaboration d'un PLU, entre 25 000 et 50 000 euros en moyenne. Si les collectivités doivent se conformer au droit, la loi doit prendre en compte leurs spécificités et leurs moyens. À cet égard, les difficultés soulevées par les élus locaux et par les auteurs de la proposition de loi sont révélatrices de la démarche encore descendante des relations entre l'État et les collectivités territoriales. L'article 1 articule expressément la procédure d'abrogation des cartes communales et l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Cette clarification au sein du code de l'urbanisme renforce la lisibilité du droit et peut ainsi représenter un gain de temps non négligeable pour les communes qui douteraient de la possibilité d'organiser une seule enquête publique et de procéder à une seule délibération pour les deux procédures. souvent engagées dans l'élaboration laborieuse d'un PLUi, il est inutile de leur compliquer la tâche pour une simple abrogation. Les précisions apportées par le rapporteur permettront de supprimer toute période pendant laquelle le RNU pouvait trouver à s'appliquer de manière transitoire entre les deux documents d'urbanisme. Bien que modeste, c'est un progrès par rapport à la situation actuelle.

En application de la loi « Engagement et proximité », qui leur a offert un an de répit, les 530 POS restants ont été frappés de caducité depuis le 1 janvier 2021. Certes, la disparition des POS au bénéfice des PLU est prévue depuis vingt ans. Cependant, remettons cela en perspective par rapport à la réalité du terrain : nous ne parlons plus que de 530 POS à épurer, parmi lesquels 130 se situent à un stade avancé du processus de transformation. Il n'y a donc pas eu d'inertie des élus locaux en la matière. Pourquoi leur refuser une souplesse, limitée dans le temps, dans un contexte de crise sanitaire et de changement d'équipes municipales ? Nous sommes persuadés que la contrainte ne crée pas d'adhésion naturelle à des projets de territoire élaborés hâtivement. Bien au contraire, il arrive qu'elle provoque des conflits qui n'existaient pas auparavant. Laissons le temps aux collectivités de construire cette adhésion, d'élaborer un document d'urbanisme de qualité permettant de répondre au développement économique local, à la sauvegarde des activités agricoles, à la préservation de la biodiversité ou à la qualité de l'habitat. Nous souscrivons donc à la démarche équilibrée du rapporteur, qui vise à temporiser les effets de la caducité des POS par l'introduction de trois aménagements à l'application du RNU permettant aux communes de continuer à préserver l'intérêt communal. Il n'est pas question d'exonérer les communes concernées de leurs obligations légales, mais simplement de leur laisser une période d'adaptation, inférieure à deux ans, le temps d'achever leur document d'urbanisme. Nous connaissons votre position, madame la ministre, sur la proposition de loi, et je ne me fais pas d'illusions quant à son adoption définitive. Néanmoins, nous espérons que le Gouvernement apportera des solutions concrètes, comme cela a été envisagé en commission. Les collectivités, majoritairement rurales, dont le processus de transformation du POS en PLU ou en PLUi est à la peine, doivent être accompagnées. L'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pourrait mettre à disposition ses compétences.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à combler un vide juridique concernant la procédure d'abrogation des cartes communales, qui n'est aujourd'hui pas explicitement prévue par le code de l'urbanisme. Il s'agit donc d'un texte utile et pragmatique, et nous remercions notre collègue Rémy Pointereau de cette initiative. Je tue d'emblée tout suspense en disant que nous voterons cette proposition de loi ... à charge de revanche La procédure définie par le texte permet judicieusement le parallélisme des formes en adossant cette procédure à celle de l'adoption d'un PLU, afin de gagner du temps et d'éviter des surcoûts.

Sur le plan de la réglementation, il est vrai que les documents d'urbanisme ont beaucoup évolué depuis la loi SRU, pour tenir compte des enjeux urbains tels que la lutte contre l'étalement urbain, l'exigence de non-artificialisation, la préservation de l'environnement et du vivant. Ce renforcement des normes et des études n'est pas, à notre sens, du « superflu coûteux ». C'est en effet utile pour atteindre les objectifs de transition et de meilleure préservation des sols. Ainsi, alors que l'équivalent d'un département disparaît tous les sept ans du fait de l'urbanisation, renforcer les objectifs et les normes nous apparaît incontournable, à l'image du « zéro artificialisation nette » prévu à l'horizon 2050. Les documents d'urbanisme sont des outils essentiels pour atteindre ces objectifs et, dans ce cadre, le renforcement des obligations de contenu nous semble aller dans le bon sens, celui de l'intérêt général.

de leur territoire. Il faut par ailleurs, même si ce n'est pas directement l'objet de cette proposition de loi, reconnaître que les évolutions auxquelles sont confrontées les collectivités tiennent beaucoup au changement d'échelle de l'exercice de la compétence « urbanisme un transfert difficile prévu par l'article 136 de la loi ALUR. Nous avions, à l'époque, formulé un certain nombre de réserves sur ce transfert automatique qui dessaisissait les communes d'un élément important dans la définition de leur projet politique. Un transfert d'autant moins opportun qu'il s'articulait avec la construction d'intercommunalités forcées, ce qui n'est pas favorable à l'émergence d'un projet urbain collectivement défini et partagé. Nous avions ainsi estimé que ce transfert de compétence venait dessaisir encore davantage les élus communaux des capacités concrètes de porter le projet politique pour lequel ils avaient été élus, participant ainsi à la vague de dévitalisation des communes et de la démocratie de proximité. Ces constructions intercommunales, réalisées parfois en dépit des volontés communales, expliquent à nos yeux pour beaucoup les retards pris dans l'élaboration des PLU et des PLUi.

et de maîtrise de leur territoire. La difficulté des collectivités à faire face à la construction de nouveaux documents d'urbanisme tient donc, à la fois, à une perte d'ingénierie humaine liée à leur dévitalisation progressive, à la fin du soutien technique de l'État

au regard des enjeux de transition écologique et d'aménagement équilibré des territoires. Pour conclure, je dirai que l'esprit de décentralisation doit être maintenu. L'État doit non pas porter une vision autoritaire de l'aménagement territorial et des collectivités, mais apporter à celles-ci son soutien puissant au service de l'intérêt général

est un texte de clarification juridique et de simplification des démarches, mais aussi de bon sens à destination des élus locaux. Permettez-moi de remercier à mon tour l'auteur de cette proposition de loi et le rapporteur de la commission des affaires économiques. Loin des débats manichéens sur le droit de l'urbanisme, en particulier loin de ceux que nous avons eus sur le transfert de la compétence en matière d'urbanisme aux intercommunalités de la loi ALUR de 2014, le texte déposé, puis celui adopté par la commission, présentent des propositions d'adaptation liées à des situations locales réelles. Dans ce texte, aucun objectif en matière d'organisation locale et aucune mesure en matière de stratégie d'aménagement ne sont remis en cause. Certains pourront éventuellement le regretter, mais la disparition des POS, la transformation des cartes communales et le transfert de la compétence aux ne sont pas remis en question. Vingt ans après la loi SRU, six ans après la loi ALUR, leurs dispositions sont appliquées, bon gré mal gré, par les territoires. Ce mouvement long est en passe d'aboutir, puisque plus de la moitié des communes françaises appartiennent à un EPCI désormais compétent en matière d'urbanisme ; plus de 18 000 PLU ont été élaborés et il restait à peine 530 POS au 31 décembre dernier. Madame la ministre, cette proposition de loi ne revient pas sur les réformes passées. Elle n'est pas non plus conservatrice. Elle a pour objectif d'accompagner les communes et les élus locaux dans cette dernière mutation.

dans le code de l'urbanisme, et un droit mou, par la jurisprudence et les instructions données aux préfets ; mouvante, parce que les lois changent souvent

Les élus locaux, on le sait bien, font leur maximum, mais reconnaissons qu'un peu de clarification et surtout d'accompagnement de la part des services de l'État ne seront jamais de trop. de loi, son article 1 apporte des précisions utiles sur la période de transition au moment du passage d'une carte communale à un PLU ou à un PLUi, et fixe une procédure plus efficace et plus lisible. S'il existe des règles ou des instructions, comme l'a rappelé le Gouvernement devant la commission, elles ne sont pas assez sûres et connues ; ce texte permet de les fixer et d'encadrer la transition. Cet article simplifie aussi certaines démarches, en limitant le nombre d'enquêtes publiques qui ont naturellement trait au même sujet. Pour l'article 2, le rapporteur a largement tenu compte de la nouvelle situation du droit après le 1 janvier de cette année. Il est proposé une boîte à outils de quelques dérogations pour les 530 communes restantes cela représente à peine 5 communes par département. Mieux vaut les aider à transformer leurs documents d'urbanisme que les braquer. Ce sera au profit de tous et, en particulier, des habitants de ces communes. Avant de conclure, madame la ministre, j'aimerais vous interpeller sur votre futur projet de loi dit « 4D ». Nous n'en connaissons encore ni toutes les mesures ni tous les détails néanmoins, prenez garde à ne pas bousculer, une fois encore, l'organisation locale en matière d'urbanisme : inutile de créer de nouveaux transferts et de nouveaux délais Il serait au contraire préférable de renforcer l'ingénierie de l'État à l'échelle départementale, pour accompagner au mieux les élus locaux. Pourriez-vous nous donner vos ambitions en la matière, en particulier vos axes de réflexion contenus dans le projet de loi 4D ?

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi a deux objectifs : expliciter le droit en matière d'abrogation des cartes communales et accorder deux ans supplémentaires aux communes n'ayant pas achevé leur transition du POS au PLU ou au PLUi au 31 décembre 2020. Quelque 530 communes en France seraient concernées par cette dernière problématique, soit environ 5 communes par département qui se retrouvent dans un état de flou juridique depuis le 1 janvier 2021, date à laquelle les POS sont devenus caducs. Il est donc tout à fait préjudiciable que l'État ait refusé de se saisir du sujet plus tôt, estimant que le droit actuel fournissait déjà des solutions. La situation aurait pu être régularisée avant la date limite de caducité, ce qui aurait évité à ces petites communes de se retrouver dans une situation difficile, sans les documents d'urbanisme qui leur permettaient de planifier leur développement. En premier lieu, on peut s'interroger légitimement sur les raisons qui expliquent ces difficultés à passer du POS au PLU ou au PLUi, difficultés qui n'ont rien à voir avec une quelconque négligence. Comme j'ai pu le souligner en commission, je maintiens que lorsqu'une petite commune appartient à une intercommunalité de taille importante, la prise en compte de ses propres intérêts peut être en soi un sujet de discussion serré. Nous abordons ici la liberté d'administration des communes : si le nouveau document d'urbanisme ne répond pas, en matière d'aménagement du territoire, aux besoins de ces communes souvent situées dans des territoires fragiles, il est compréhensible qu'elles aient besoin de temps pour affiner son élaboration. Était-il possible de fournir à ces communes les moyens nécessaires en ingénierie et en finances pour tenir les délais ? Sans doute, mais cela n'a pas été anticipé, d'où la situation où elles se trouvent aujourd'hui. Notre rôle en tant qu'élus des territoires est de nous montrer à l'écoute de ces difficultés et d'y apporter une réponse. En l'absence de tout document d'urbanisme, ces communes reviennent au RNU. Je sais, madame la ministre, que vous jugez cette solution tout à fait applicable ; vous rappelez que quelques maires ruraux de votre connaissance souhaitent conserver ce régime d'urbanisme.

C'est un régime restrictif où les situations se règlent au cas par cas, selon la libre appréciation des directeurs départementaux des territoires. Le manque de transparence est donc total, et le risque de voir des prédateurs fonciers lésés par les précédents documents d'urbanisme devenus caducs tenter d'exploiter les ambiguïtés permises par le retour au RNU est réel. Un retour à ce dispositif va à l'encontre de la lutte contre l'artificialisation des sols et n'assure pas aux communes des conditions de développement semblables à celles qui étaient prévues dans les POS. Le Sénat s'est vu contraint d'examiner le présent texte après la date limite de caducité ; les auditions menées par le rapporteur ont permis de constater que ce vide juridique entraînait la perte de la maîtrise foncière et du droit de préemption urbain, ainsi qu'un risque de blocage de certains projets à cause du retour au RNU. Une réécriture complète de l'article 2 de la proposition de loi a donc été proposée, de manière à atténuer les conséquences de la caducité des POS par la mise à la disposition des maires des communes concernées d'une boîte à outils applicable jusqu'à l'adoption du nouveau PLU ou PLUi, et jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard. Le texte de la commission prévoit également de créer un droit de proposition des maires : ils pourraient solliciter du préfet l'usage de son pouvoir de dérogation aux règles du RNU pour des projets qui auraient été compatibles avec le POS antérieur, mais ne le sont pas avec le RNU. Le Gouvernement s'est pourtant montré opposé à ces mesures transitoires, arguant que, sur les 530 communes évoquées, 160 communes seulement se situaient à l'arrêt du projet de PLUi et 200 autres à un stade d'avancement très faible, tandis que 130 communes revenues au RNU allaient pouvoir approuver rapidement leur PLUi. Sur le droit de proposition, madame la ministre, vous avez émis un avis défavorable au motif que le maire restait l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sous la seule réserve de recueillir l'avis conforme du préfet. Malheureusement, votre argumentaire ne fonctionne réellement que dans le cas où les deux parties sont d'accord. Même si le maire reste libre de ne pas suivre les conclusions du préfet, il n'est pas toujours évident d'aller contre l'avis de l'administration. Pour ces 360 communes, madame la ministre, vous avez proposé en commission d'écrire à tous les préfets pour vous faire remonter avec précision pourquoi certaines communes ou intercommunalités connaissent des situations de blocage. Vous proposez enfin d'accompagner au plus près ces collectivités,

le sujet est de la même importance pour une agglomération ou pour une petite commune, et toutes deux sont utiles à nos territoires. Le groupe socialiste confirmera donc le vote favorable qu'il a eu en commission sur cette proposition de loi, en espérant que la navette parlementaire sur ce texte s'achèvera dans les délais de la présente législature. En effet, si tel n'était pas le

la proposition de loi de notre collègue Rémy Pointereau que nous examinons en cette fin d'après-midi va assurément dans le bon sens. Elle vient sécuriser certains vides juridiques identifiés sur nos territoires par les élus locaux, que ce soit au sein des communes ou des EPCI. Nous l'avons suffisamment dit ici : il existe encore des difficultés, notamment dans de petites communes rurales et de petits EPCI, même si la couverture des PLU et des PLUi progresse sur le territoire hexagonal.

Dans le premier cas, la date limite, repoussée à plusieurs reprises, est désormais dépassée depuis la fin du mois de décembre dernier. Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de notre examen de ce texte en commission la semaine passée, les ralentissements ont

texte apporte donc des réponses pratiques et réalisables. Je salue ce que nous appelons la « procédure combinée » et son approfondissement. Elle me paraît être logique et pragmatique. Comme j'ai pu également le dire lors du débat en commission, l'article 2 de cette proposition de loi et la boîte à outils qui y est développée sont les bienvenues pour les 530 communes concernées. Les possibilités qui sont données aux maires dans le cadre des autorisations d'urbanisme et des dérogations aux règles du RNU auront des finalités concrètes. Le couple maire-préfet serait

D'autres objectifs du droit de préemption urbain sont quant à eux impossibles à mobiliser, ce qui risque de susciter des difficultés pour les communes concernées.

détaillées à l'article 2. Il me paraît essentiel qu'au-delà du 31 décembre 2022 les transitions aient pu être effectuées et que les effets négatifs des situations actuelles soient définitivement derrière nous. Là encore, nous devons rester attentifs et accompagner ces communes. Le rôle des préfets et des maires demeure central. Ils doivent oeuvrer de concert : c'est un gage de solutions pour nos territoires, c'est aussi l'esprit de ce texte. Pour conclure, je suis amené à constater sur le terrain que les politiques d'urbanisme ne sont pas toujours adaptées aux territoires ruraux. Si je conviens qu'il faut lutter contre l'artificialisation des terres et l'étalement urbain, il ne faut pas pour autant exclure les territoires ruraux de leur développement urbanistique. Les politiques actuelles sont quelquefois trop restrictives : il devient parfois impossible de proposer des terrains à bâtir aux enfants de nos villages. Leur développement, indispensable,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous partageons l'objectif tout à fait louable de cette proposition de loi, qui permet de mieux accompagner la transition des documents d'urbanisme communaux vers les PLU et PLUi. ces règlements a fait l'objet d'un certain nombre de réformes importantes depuis les années 2000 ; je n'en referai pas l'historique. Ce texte s'attelle d'abord à une simplification et à une clarification bienvenues

Il convient donc de clarifier et d'expliciter le droit et de lever des contraintes inutiles, pour ne plus exposer des communes à une potentielle insécurité juridique. Ce sont surtout les plus petites d'entre elles qui peuvent être mises à mal, celles qui sont peu accompagnées dans ces évolutions procédurales et qui n'ont pas les moyens humains et financiers d'y faire face d'entre elles, je dirais plutôt qu'elles n'ont plus ces moyens. En ce sens, l'article 1 nous paraît tout à fait pertinent : il fixe dans la loi la procédure applicable, qui permet de sécuriser juridiquement ces communes et d'apporter aux élus locaux des outils clairs et efficaces pour davantage de prévisibilité. Il apporte notamment une souplesse accrue aux collectivités et aux intercommunalités, lorsque l'abrogation d'une carte communale intervient au profit de l'approbation d'un PLUi, et prévoit ainsi une procédure combinée d'abrogation de la carte communale et d'approbation du PLUi PLUi une enquête publique unique et une seule délibération finale. Voilà le plus important ! Nous saluons le renforcement par la commission de cette procédure combinée, qui sera prévue dès la délibération initiale de prescription. Cela tend à éviter tout décalage entre l'abrogation des cartes et la mise en application du PLUi, et permet d'éviter la mise en application temporaire du RNU. L'article 2 initial, qui reportait de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, la date de caducité des POS nous posait davantage question l'argument selon lequel la crise sanitaire et la période de confinement auraient empêché l'avancée de certaines communes sur leur document d'urbanisme peut s'entendre, mais notons que cela fait tout de même vingt ans que la disparition des POS doit être actée. Un an supplémentaire nous paraissait largement suffisant pour laisser les 530 communes concernées faire aboutir leur PLUi. Comme nous l'avons vu en commission, ce délai supplémentaire est inopérant puisque la caducité a été actée depuis le 1 janvier. La commission a donc proposé d'apporter des dérogations facultatives, ciblées et encadrées dans le temps aux maires des communes concernées par la caducité, en se basant sur un dialogue renforcé entre le maire et le préfet.

Nous restons tout de même vigilants : ces dérogations doivent être suffisamment cadrées et ne sauraient permettre de revenir temporairement sur des réglementations nécessaires pour la protection des paysages et de la biodiversité, en lien avec l'artificialisation des sols ou la protection du littoral. garde à ce que ce délai supplémentaire ne soit pas utilisé comme un moyen de déroger à l'application de documents d'urbanisme qui s'imposeront aux futurs PLU ou PLUi. Je pense notamment aux SCoT. Merci, madame la ministre, monsieur le rapporteur, de nous apporter des éléments sur ce point. Pour conclure mon explication au nom du groupe écologiste, nous voterons pour ce texte qui permet globalement de clarifier le droit et apporte des outils utiles aux élus locaux.

le transfert au niveau communal de la compétence en matière d'urbanisme, en 1983, plusieurs réformes sont intervenues pour encadrer l'action des collectivités en la matière. Avec les lois SRU et ALUR, les documents d'urbanisme sont devenus de véritables instruments d'aménagement et de cohésion des territoires, intégrant des objectifs de contrôle de l'étalement urbain, de mixité sociale, ou encore, plus récemment, de lutte contre le changement climatique. Avec la complexité croissante des règles en matière d'urbanisme, aggravée dans certaines collectivités par le manque d'ingénierie et de moyens financiers, les maires et les présidents d'intercommunalité peuvent rencontrer des difficultés dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Aussi, la proposition de loi que nous examinons entend épauler ces collectivités face à ces difficultés. Il est question, d'une part, à l'article 1, de clarifier et d'expliciter la procédure applicable applicable en matière d'abrogation des cartes communales, et, d'autre part, à l'article 2, de répondre aux inquiétudes suscitées par la disparition des POS. En commission, nous avons salué la volonté de sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales portée à l'article 1 par les auteurs de cette proposition de loi. Mais si le droit se doit d'être lisible, la codification proposée ne nous a toutefois pas semblé nécessaire. jurisprudence, reprise par de nombreuses instructions ministérielles et confirmée dans la pratique, démontre que les solutions existent et sont opérationnelles. Or, en matière de codification, le mieux s'avère parfois être l'ennemi du bien. Aussi, notre crainte est que l'introduction de nouvelles dispositions dans le code de l'urbanisme génère de nouveaux contentieux et qu'elle nuise davantage à la lisibilité du droit En revanche, les auteurs de la proposition de loi ont relevé à juste titre l'existence d'un vide juridique durant la courte période qui sépare le moment de l'abrogation de la carte communale de celui de l'entrée en vigueur du PLU. Si le texte a le mérite de proposer une solution pour combler ce vide juridique, la voie législative ne nous semble pas la plus appropriée, en raison notamment du temps qui serait nécessaire pour une mise en oeuvre effective de cette solution. En conséquence, nous avons choisi en commission de faire confiance à Mme la ministre, qui s'est engagée à apporter une solution à cette situation par la voie réglementaire. Une instruction claire rappelant les règles d'abrogation des doit par ailleurs être envoyée aux préfets. Nous nous sommes montrés plus sceptiques en ce qui concerne l'article 2, qui reportait à l'origine de deux ans la date de la date de caducité des POS. Il s'agissait de tenir compte du retard pris par certaines communes dans l'élaboration de leur PLU, notamment du fait de la crise sanitaire. Si nous comprenons l'inquiétude suscitée par cette caducité, un tel report nous aurait semblé inéquitable par rapport aux communes qui ont accéléré l'adoption de leurs documents d'urbanisme et ont tenu les délais. Par ailleurs, le principe de non-rétroactivité de la loi s'opposait à ce que l'on revienne sur la caducité des POS intervenue au 1 janvier 2021. Enfin, un énième report ne nous a pas semblé opportun, alors qu'il ne reste que 530 communes concernées et qu'une grande partie d'entre elles sont en train de terminer l'élaboration de leur document d'urbanisme. Cet article a toutefois été complètement réécrit en commission. S'il n'y est plus question de report de la caducité des POS, la rédaction proposée revient par des voies de contournement aux mêmes finalités. En conséquence, cette nouvelle rédaction ne modifie pas notre notre regard sur l'objet de cette mesure. Conscients toutefois des difficultés que peuvent rencontrer certains élus en matière d'urbanisme, nous observons avec bienveillance la démarche portée par ce texte. Nous ne pouvons néanmoins totalement y souscrire, puisque les solutions qui y sont proposées s'avèrent déjà satisfaites ou trouveront une traduction plus rapide et plus efficace par la voie réglementaire. Aussi, comme Mme la ministre a entendu les difficultés exprimées et s'est engagée à y répondre, nous choisirons de nous abstenir.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi que j'ai déposée, avec l'appui de plus de 80 sénatrices et sénateurs, le 18 décembre 2019. Sans vouloir retracer la genèse de cette initiative, je souhaite tout de même indiquer qu'elle émane du terrain, de nos collègues élus locaux qui sont excédés par les changements permanents du cadre juridique des règles et documents d'urbanisme locaux. Cette proposition de loi, qui aurait pu se transformer en simple amendement, reflète parfaitement le manque d'information que subissent nos collègues de terrain. Dès l'automne 2019, j'ai été interpellé par le président d'une communauté de communes de mon département et par plusieurs maires ; ils m'ont fait part de leur incompréhension de voir les cartes communales abrogées dès lors que la communauté de communes lance une enquête publique dans le cadre de l'élaboration de son PLUi, avant même que celui-ci soit validé ! Il n'est pas question d'une courte période

Malheureusement, aucune loi ne précise comment s'opère cette transition. Le rapport de notre collègue Jean-Baptiste Blanc, que je félicite au passage pour son travail et son investissement sur le sujet, indique qu'en l'absence d'informations claires,

l'abrogation de la carte prendra effet dès lors que le nouveau document, tel qu'un PLUi, entre véritablement en vigueur. C'est une mesure pragmatique et de bon sens qui comble un vide juridique pour faciliter le travail de nos élus locaux.

que je ne suis pas le seul à avoir été saisi de la question, qui a été posée dans de nombreux départements. Comme vous le savez, la loi ALUR a instauré un principe de caducité des POS qui a connu- soyons honnêtes ! -plusieurs assouplissements en matière de délais. résulte d'ailleurs d'une initiative sénatoriale, puisqu'un report d'un an, soit jusqu'au 31 décembre dernier, avait été obtenu lors de l'examen du projet de loi « Engagement et proximité ». Malheureusement, 536 communes n'ont pas eu le temps de finaliser leur PLUi avant la caducité du POS. Cela s'explique parfois par des raisons financières un PLU coûte en moyenne entre 25 000 et 50 000 euros ; une commune n'allait pas investir une telle somme alors qu'un PLUi allait bientôt Mon idée de départ était de faire la même proposition que pour les cartes communales : préciser que l'abrogation du POS ne prendrait effet qu'à partir du moment où le PLUi entrerait en vigueur, afin d'éviter de revenir au RNU. Malheureusement, le délai du 31 décembre étant passé, le dispositif que j'avais proposé n'est plus viable. Pour une collectivité, retomber sous le régime du RNU entraîne d'importantes conséquences : perte du droit de préemption urbain ; exigence d'un avis conforme préalable du préfet sur les autorisations délivrées par le maire au nom de l'État ; restrictions de construction pour les zones non urbanisées.

Je sais, madame la ministre, que vous êtes opposée à ce dispositif, pourtant de bon sens, et que vous considérez- vous l'avez dit en commission -que les communes frappées

Madame la ministre, vous avez été élue locale, maire, présidente de communauté de communes. Vous ne pouvez donc pas aujourd'hui ignorer les difficultés des maires, qu'ils soient 536 ou même une dizaine. Le Sénat, maison des territoires et des élus, s'honore et s'oblige à leur trouver des solutions. En conclusion, je remercie la commission des affaires économiques et son rapporteur, Jean-Baptiste Blanc, d'avoir trouvé des solutions concrètes

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, la proposition de loi visant à sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales dans le cadre d'une approbation d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et à reporter la caducité des plans d'occupation des sols (POS). L'ordre

Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

je me réjouis que ce débat puisse avoir lieu au sein de notre hémicycle, tant ce sujet suscite à la fois de vives inquiétudes et des récupérations politiques de toutes sortes. Il s'agit d'un sujet sensible- c'est heureux qu'il le soit et il faut

Notre pays peut s'enorgueillir d'être une terre d'accueil, et c'est afin qu'il puisse le demeurer que nous devons être fermes avec ceux qui chercheraient à dévoyer sa politique. Il faut parfois le rappeler, lorsque nous évoquons les mineurs non accompagnés (MNA), nous parlons avant tout de vies brisées et d'enfants déracinés. Oui, tout enfant privé de son milieu familial, sur notre sol, mérite notre protection. certains individus sans vergogne cherchent à bénéficier des moyens qui ne leur sont pas réservés, et nuisent ainsi à la qualité de prise en charge de ces mineurs en grande difficulté. Cet accueil, qui est d'abord le reflet d'un drame humain, a aussi un coût, 2 milliards d'euros par an, et l'Assemblée des départements de France (ADF) nous alerte sur le fait que près de 70 % de prétendus mineurs ne le sont pas en réalité. Je vous laisse faire le calcul Pour pouvoir être à la hauteur de notre idéal, nous devons, sans relâche et de manière concomitante, lutter contre les réseaux qui exploitent cette misère humaine. Certains témoignages au sein des établissements En effet, il arrive que le personnel voie plusieurs individus se présenter devant eux avec exactement le même certificat de naissance. sans scrupules, avec l'aide de passeurs, cherchent à être identifiés comme mineurs et connaissent parfaitement notre système administratif et ses failles. Nos départements sont débordés et les coûts imposés sont très supérieurs à la compensation accordée par l'État. Sous l'actuelle présidence, et après des heures de négociation, la participation de l'État est passée de 12 % à 14 %, alors que ces mineurs étaient 4 000 en 2010, contre près de 40 000 aujourd'hui. évoqué des coûts « imposés », car le Gouvernement ne fait rien pour y remédier. En effet, certains départements, par idéologie ou par posture politicienne, fragilisent l'ensemble de notre politique d'accueil. La gestion des flux migratoires est une compétence non pas départementale, mais bien régalienne. Il revient désormais à l'État de porter ses responsabilités. C'est bien l'État qui rend possible qu'un tiers des départements se refusent à renseigner un fichier national recensant les demandes de prise en charge, et permettant ainsi de lutter contre les demandes répétitives et abusives.

Dans un article publié dans le 7 novembre dernier, le ministre de l'intérieur se désolait qu'il n'y ait pas d'obligation à remplir ce fichier.

handicapent sciemment notre politique d'accueil, et je crains que l'incitation financière née du décret du 23 juin 2020 ne soit pas suffisante. Une nouvelle fois, il s'agit de décourager des individus qui cherchent à bénéficier d'aides dues à des mineurs en détresse. Pour y parvenir, puisque ces personnes se présentent sous de faux papiers- quand elles ne se présentent pas sans papier -, nous devons pouvoir recourir aux tests osseux qui, bien qu'ils ne soient pas infaillibles, contribuent à établir un faisceau d'indices dont nous ne pouvons pas nous passer en la matière. Prenons le temps, à cet égard, de préciser qu'il s'agit d'une simple radiographie, et que celle-ci peut être refusée. En somme, nous devons nous préoccuper de la véracité de la situation du demandant. Il importe de constater sa minorité comme son isolement. En la matière, nous devons nous donner beaucoup plus de moyens. Il y a peu, j'ai eu à solliciter la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la étaient débordés, alors même qu'il s'agissait en l'espèce d'une ressortissante de bonne foi. Faisant ce constat, je ne pouvais que m'interroger, non sans perplexité, sur le suivi susceptible d'être réservé au demandeur dont la majorité avait été établie Cette tentation, que certains départements font naître, fait le jeu de réseaux mafieux. En effet, ceux qui sont déboutés, bien qu'étant en situation irrégulière, ne résident pas moins sur le sol français et devront, dans l'attente d'un éloignement, subvenir à leurs besoins.

Les réseaux sont alors doublement gagnants, et j'espère ne pas être le seul à ne pas m'y résoudre. Car cette générosité d'apparat, facile à tenir en discours, nuit à notre capacité d'accueil. Ces enfants- car nous parlons bien d'enfants ! -doivent pouvoir bénéficier d'une formation, être logés et suivis. Cela représente un coût estimé à 50 000 euros par an et par enfant, sans compter d'éventuels frais de santé.

Nous ne pouvons laisser de faux mineurs user de notre générosité et ainsi grever l'assistance à ces jeunes au parcours déjà si difficile.

victimes d'enfermement aux frontières, dans les centres de rétention administration et dans les zones d'attente, avant d'être bien souvent criminalisés ou pointés du doigt ... Je vous le redis avec force : nous ne pouvons pas traiter ces mineurs étrangers autrement que comme nos propres enfants. L'intérêt supérieur de l'enfant et la protection de l'enfance doivent toujours

déjà en réalité. Il relève de nos obligations internationales et de notre droit interne de mettre à l'abri toute personne se déclarant mineure.

d'asile (Ceseda), pour que le critère de suivi d'une formation à l'admission au titre de séjour soit élargi aux formations d'enseignement général. Enfin, la proposition n° 30

dans la prise en charge des mineurs non accompagnés, en tout cas de ceux qui se déclarent comme tels. Il insistait en particulier sur le manque de pilotage et d'organisation interministériels, et soulignait même des fragilités.

au sein de l'État qu'entre l'État et les départements.

Face à l'augmentation massive du nombre de MNA étrangers, qui a triplé entre 2016 et 2018, même si cela va un peu mieux maintenant, les services départementaux doivent s'organiser dans l'urgence sans les moyens et les structures adaptées. de vue budgétaire, les dépenses ont considérablement augmenté. À titre d'exemple, le département des Côtes-d'Armor dépensait 2,5 millions d'euros pour la prise en charge des mineurs non accompagnés en 2016, contre 8 millions d'euros Certes, il reçoit des aides de l'État, mais celles-ci sont loin de compenser toutes les dépenses. En 2019, l'État budgétait ainsi seulement 141 millions d'euros, alors que le coût évalué par l'ADF était- je le rappelle -de 2 milliards d'euros. C'est un gouffre financier pour les départements, qui s'ajoute d'ailleurs à la non-compensation croissante des allocations individuelles de solidarité. Chaque département se voit imposer chaque année par l'État un pourcentage de MNA à accueillir, se révèlent parfois, au terme d'une procédure d'évaluation ou même au cours de leur prise en charge, être des majeurs. L'État laisse les collectivités gérer seules les conséquences de son manque de courage politique. Une fois de plus, il est aux abonnés absents La question des MNA est liée à la politique migratoire, monsieur le secrétaire d'État. C'est donc bien une prérogative régalienne. Cerise sur le gâteau, le Gouvernement vient de décider unilatéralement d'interdire aux départements d'héberger les MNA dans des hôtels, tout cela sans proposer de solution de remplacement. D'ailleurs, il n'en existe pas. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement a-t-il l'intention de prendre sa part de responsabilité dans la gestion du flux migratoire, afin de désengorger les demandes d'accueil et d'accompagnement de ces jeunes et d'assumer ainsi ses responsabilités ? Va-t-il enfin soutenir efficacement les conseils départementaux en leur donnant les moyens nécessaires pour accueillir ces mineurs non accompagnés ?

proposer d'autres solutions, et même un encadrement strict dans le temps sur les modalités d'accompagnement et le type d'hôtel,

j'ai pu m'entretenir avec une famille accueillant trois mineurs isolés étrangers. Deux d'entre eux, jeunes gens de nationalité pakistanaise, venaient du foyer où était hébergé l'auteur de l'attentat. Je dois dire que plusieurs points m'ont interpellé au cours de mes échanges avec cette famille d'accueil. Ces deux jeunes mineurs considéraient de bonne foi le blasphème comme un crime. Ils approuvaient même l'attentat qui venait d'être commis. Le couple qui les accueille a pris le parti, contre l'avis des éducateurs, de leur enlever quelque temps après l'attentat leurs téléphones, grâce auxquels ils entretenaient des liens avec d'autres personnes partageant cette opinion. Les deux mineurs ont également été entendus par des gendarmes. J'ai été surpris de constater qu'aucun suivi éducatif ou pédagogique ne leur avait été apporté dans leur foyer d'origine. Il n'y a pas de cours d'éducation civique leur permettant de s'intégrer en acquérant les valeurs de la Nation française En fait, ils viennent avec leur culture et ignorent la nôtre. À ce titre, l'insertion en lieu de vie, plutôt qu'en foyer, semble être une bien meilleure solution. Les lieux de vie sont sous-utilisés, et nos départements manquent de moyens pour réaliser ces accueils dans de bonnes conditions. Dans le témoignage que j'ai recueilli, les accueillants m'ont affirmé que ces jeunes gardaient des contacts réguliers avec leur famille. Dans ce cas, si l'on connaît les parents, si l'on peut les identifier, pourquoi ces jeunes restent-ils en France ? Enfin, les passeurs sont souvent connus dans le cas des mineurs non accompagnés ; c'était le cas pour ces deux jeunes. Ces gens utilisent la misère du monde. C'est inadmissible

En effet, les délais de traitement des recours de reconnaissance de minorité auprès d'un juge peuvent varier de six à vingt-quatre mois, et certains jeunes arrivent à majorité avant d'obtenir une réponse. Par ailleurs, on note de grandes disparités territoriales : dans certains départements, l'évaluation de ces mineurs ne va durer qu'un seul jour ; dans d'autres, ils seront placés à l'hôtel pendant plus de six mois.

qui est problématique en plein hiver et en pleine pandémie. De ce fait, non seulement il apparaît urgent d'appliquer immédiatement la présomption de minorité pour ces jeunes en recours, mais il convient aussi d'aller au-delà et de tout simplement prendre en compte leur vulnérabilité pour qu'ils aient accès à une réelle prise en charge Les associations qui pallient ces carences ne peuvent pas remplacer à elles seules l'État. Quand celui-ci prendra-t-il ses responsabilités ? La parole

Mohamed Soilihi. Monsieur le secrétaire d'État, lorsqu'elle porte sur Mayotte, la question des mineurs non accompagnés déborde largement le champ de la politique de l'aide sociale à l'enfance ou du secteur associatif. La situation du 101 département reste en effet singulière sur le territoire national. Je ne peux pas éluder en disant cela les événements très graves qui se produisent sur le sol mahorais, opposant des bandes de jeunes armés, lesquels ont très récemment tué deux mineurs. La particularité se retrouve également dans les chiffres, rappelés par le dernier rapport de la chambre régionale des comptes sur le sujet. Ainsi, plus de 4 000 MNA ont été dénombrés en 2016.

dans son rapport de 2020, justifie de cette façon le fait que ce département ne soit pas pris en compte dans les données nationales qu'elle utilise. Cette spécificité est aussi celle de la situation géographique de Mayotte, qui se traduit par une pression migratoire insupportable depuis les Comores, par l'absence de répartition entre départements de la prise en charge des MNA se trouvant sur le sol mahorais, lesquels sont livrés à une grande précarité et à toutes les vulnérabilités.

À ce titre, quel bilan pouvez-vous dresser de l'action de l'État en appui du département ? Je pense notamment à la convention de 2017 relative aux concours en faveur de l'ASE. Dans la continuité, quelles actions sont-elles envisagées pour traiter cette réelle difficulté de prise en charge des MNA dans notre département ?

de cette dotation exceptionnelle. Vous le savez, lors de ma venue, j'ai apporté un concours financier exceptionnel de 2 millions d'euros à destination non pas du conseil départemental, mais directement des associations qui agissent auprès des enfants à Mayotte. Il s'agit de les aider à créer des places supplémentaires et à mettre en place des dispositifs de prévention spécialisée. J'ai par ailleurs tendu la main au président du conseil départemental,

Mme Nathalie Delattre. Monsieur le secrétaire d'État, depuis deux ans, la quiétude et la sérénité qui caractérisaient notre belle ville de Bordeaux sont perturbées par l'afflux massif de jeunes étrangers isolés. Ils sont livrés à eux-mêmes, errant dans le centre-ville et devenant ainsi les proies idéales de réseaux de traite d'êtres humains. La hausse des violences est sans précédent : vols à l'arrachée, cambriolages, agressions, trafic de stupéfiants et d'armes sont devenus monnaie courante. Pour la préfecture, plus de 40 % de la délinquance des mineurs à Bordeaux seraient le fait de ces mineurs non accompagnés eux ont d'ores et déjà été pris en charge par le département, mais au moins 200 posent encore problème. Pourtant, une trentaine seulement seraient réellement âgés de moins de 18 ans.

Nous devons faire ici l'aveu de l'échec de notre politique d'évaluation de l'âge de ces étrangers, malgré quelques coopérations fructueuses, mais trop lourdes, avec l'Espagne. Il faut mettre un terme aux polémiques stériles qui surgissent de toutes parts et nous empêchent d'avancer. Sur les tests osseux, l'avis du Conseil constitutionnel de 2019 aurait dû mettre un terme à certaines controverses injustifiées, d'autant que ces examens radiologiques, sous-exploités, sont la seule solution pour régler l'épineuse question de la présomption de minorité. n'est-il pas systématique lorsqu'un jeune migrant souhaite contester la décision du département devant un juge pour enfants, seul habilité à statuer définitivement sur l'âge

Annick Jacquemet. Monsieur le secrétaire d'État, après une dizaine d'années d'augmentation exponentielle du nombre de MNA accueillis dans nos départements, le nombre de jeunes mineurs étrangers semble se stabiliser. Il est temps maintenant de faire fonctionner correctement le système. Les départements réclament de la cohérence entre les actions de chaque intervenant : la justice, l'État et les collectivités. Le système souffre en effet d'un parcours en deux étapes qui crée de fausses espérances pour les jeunes et des coûts indus importants pour les collectivités. J'attire votre attention, monsieur le secrétaire d'État, sur ce qui pourrait constituer une incohérence dans la mise en oeuvre de notre politique publique. accueil du jeune par la protection de l'enfance. Le doute sur la minorité profite à l'intéressé et l'état civil est rarement reconstitué. Les jeunes bénéficient alors d'un système très généreux qui va les accueillir, les former et les accompagner

Il apparaît donc nécessaire de déterminer très rapidement, dès l'arrivée des MNA en France, leurs chances d'y séjourner durablement, avant qu'ils ne prennent racine dans notre pays sans espoir de pouvoir y rester. Nous avons évoqué le cas du jeune Traoré. Le fichier AEM est très efficace. Il apporte toutes les garanties au jeune en matière de recours devant le juge des enfants. Son utilisation doit être généralisée à l'ensemble des départements. également nécessaire de déterminer très rapidement les chances des mineurs de rester durablement dans notre pays, en rendant obligatoire le dépôt anticipé d'une demande de titre de séjour

77 MNA ont été mis en cause dans 254 infractions. Systématiquement, quand ils passent devant la justice, ils sont remis en liberté à la charge du département, même lorsqu'ils sont jeunes majeurs.

mais il ne permet pas toujours un accompagnement social débouchant sur une réelle intégration et insertion professionnelle. Ainsi, depuis 2015, la proportion de jeunes de plus de 16 ans pris en charge mais non scolarisés a largement augmenté, malgré le souhait de la plupart d'entre eux de poursuivre leur formation

Qu'attendez-vous pour que la réponse judiciaire soit à la hauteur des préjudices moraux et financiers subis par des milliers de citoyens français ? Bien souvent, l'absence de recours aux tests osseux conduit à abandonner les poursuites et à remettre en liberté des délinquants que la police qualifie de « mijeurs » : ils se disent mineurs, mais tout le monde sait qu'ils sont majeurs.

essayer d'y remédier. Mais il faut aussi dire que notre système protège des dizaines de milliers d'enfants chaque jour qui passe. C'est l'honneur de notre pays d'avoir un tel système, l'honneur des départements d'en assumer la responsabilité, l'honneur des travailleurs sociaux

mineurs. La réforme de la clé de répartition, à laquelle je m'étais engagé, a permis de retenir comme critère démographique la population générale, et non pas les seuls jeunes de moins de 19 ans présents sur le territoire.

On constate que l'évaluation de la minorité est défaillante, cela a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui. Les conséquences sont importantes : cette fraude massive représente un coût exponentiel pour les budgets de la protection de l'enfance. En effet, l'État ne finance que la phase d'évaluation et de mise à l'abri sur une durée maximale de vingt-trois jours, alors que les mineurs non accompagnés sont confiés aux départements en moyenne au moins deux ans. Pour la collectivité européenne d'Alsace, par exemple, où les mineurs non accompagnés viennent souvent des filières mafieuses des pays de l'Est, qui ne sont pas en guerre, mais où

L'autre difficulté, c'est que nous sommes face non plus à des enfants, mais à de jeunes adultes, qui s'intègrent moins facilement à la culture française. Parce que leur insertion est plus compliquée, des phénomènes de violences, de drogues et d'addictions apparaissent dans les lieux d'accueil qui sont normalement réservés à l'enfance mineure isolée. En milieu carcéral, les établissements pénitentiaires pour mineurs observent l'émergence d'un phénomène nouveau. La violence explose ; les personnels des lieux d'incarcération pour les mineurs l'affirment : huit mineurs sur dix sont en fait majeurs. Pour sortir de cet engrenage, seul un système d'évaluation de l'âge, avec des tests osseux, que l'on a déjà évoqués, médical, centralisé, et contrôlé permettrait aux départements de revenir à leur vraie mission, celle de l'accompagnement et de l'insertion de ces jeunes de moins de 18 ans. Ma question est la suivante : au lieu de prendre le problème à la source, pour éviter aux départements d'avoir à gérer des faux mineurs illégaux qui leur coûtent très cher, pourquoi votre futur projet de loi s'attache-t-il surtout à contrôler l'action sociale des départements par les préfets ?

à ce que la réforme que j'évoquais tout à l'heure ne conduise pas à un contrôle par les préfets de l'action sociale des départements. Ce n'est pas du tout mon intention et cela n'aurait pas de sens, me

Je ne reviens pas sur la question des conditions d'évaluation, notamment sur le recours aux tests osseux. Une fois encore, je n'ai pas de souci, par principe ou par idéologie, avec les tests osseux ; je mentionne simplement les limites scientifiques de son recours. Je constate que le Conseil constitutionnel a estimé que ce n'était pas contraire à la dignité humaine, mais que cela ne peut pas être l'élément unique

Pour ma part, à l'issue de ce débat, je veux attirer votre attention sur le continuum de la protection de l'enfance, qui doit concerner les MNA, comme tous les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. En effet, ces jeunes bénéficient d'un accompagnement de l'ASE au titre du contrat jeune majeur. Or, nombre d'entre eux doivent mettre un terme à leur parcours d'insertion en raison de leur situation administrative. Alors qu'ils sont engagés dans un parcours scolaire et/ou d'apprentissage, leur majorité, faute de titre de séjour, les condamne. Les mêmes pour lesquels l'État a demandé aux conseils départementaux d'assurer la protection et la prise en charge inconditionnelle sont ensuite parfois chassés par ce même État, de manière aveugle, alors qu'ils sont bien souvent en phase d'insertion et de construction d'un nouveau projet de vie. Les services de l'ASE instruisent régulièrement une demande d'asile auprès de l'Ofpra ou d'accession à la nationalité française, lorsque cela est possible, mais se heurtent à des blocages liés bien évidemment au fait que ces jeunes MNA ne disposent souvent pas de documents d'état civil authentifiés par les services de la Bref, nous sommes dans un cadre kafkaïen, qui provoque de véritables drames humains. Ces parcours interrompus stoppent l'engagement de ces jeunes, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État. Ils mettent aussi en difficulté des entreprises qui avaient investi dans leur parcours d'apprentissage et qui se retrouvent accusées d'avoir recours au travail clandestin. Ce n'est acceptable ni pour les jeunes, ni pour les entreprises, ni pour les professionnels de l'ASE qui voient leurs missions niées, ni pour nos finances publiques, qui ont investi sur ces jeunes pour les abandonner ensuite. Dans mon département par exemple, le Cantal, plusieurs jeunes sont dans cette situation, et les réponses administratives apportées, qui confinent à l'impuissance, sont désespérantes pour tous, y compris pour notre reconquête démographique.

secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, au risque de me répéter un peu, c'est, je crois, tout le sens de ce que nous essayons de faire pour les mineurs non accompagnés, comme pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. En effet, la question de la majorité, c'est-à-dire de la fin de la prise en charge dans un certain nombre de cas par les services de l'aide sociale à l'enfance à 18 ans, soulève, s'agissant de l'aide sociale à l'enfance, à l'enfance, un certain nombre de questions, de difficultés, parfois de situations dramatiques, avec ce que l'on appelle les sorties sèches. Un certain nombre de jeunes, du jour au lendemain, ne sont plus pris en charge. dans un cas comme dans l'autre, je pense que la coopération entre l'État et les départements et ce continuum que vous évoquiez doit être mobilisée au maximum. C'est tout le sens, s'agissant de l'insertion professionnelle, de cette convention avec l'Union nationale des missions locales que j'évoquais et à laquelle nous avons adjoint une contribution financière de la part de l'État de 500 euros pour tout jeune qui ne serait pas dans un parcours d'études ou d'insertion, d'éviter justement ces fameuses sorties sèches. Je précise ici que cette mesure n'a pas vocation à se substituer à un éventuel contrat jeune majeur, ou en tout cas à l'accompagnement éducatif qui pourrait continuer à être nécessaire de la part du département.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, conclure un tel débat est une gageure, c'est évident. En tout cas mon propos, qui va relever certaines des questions qui ont été abordées, n'a pas vocation à mettre un point final, bien évidemment, mais à faire saillir quelques éléments. Le point principal par lequel je voudrais commencer, c'est la nécessité et le caractère indispensable du débat que nous avons et

doit nous interroger en tant que responsables publics. Quelles en sont les causes ? Examinons les conséquences et essayons de comprendre ce qui se passe. Ensuite, cela a été dit également, monsieur le secrétaire il s'agit là d'une compétence départementale majeure, particulièrement sensible et même emblématique de l'action sociale des départements. Pour avoir siégé pendant près de sept ans au bureau de l'Assemblée des départements de France, je puis vous assurer que l'ensemble des présidentes et présidents de départements ont à coeur de remplir cette noble mission de donner une deuxième chance à ces enfants qui ne trouvent pas toutes les chances dans leur famille. Je puis attester qu'ils y sont tous très attachés. C'est justement cela qui les amène à s'inquiéter de cette situation de dégradation.

du débat. Nous avons affaire maintenant à un phénomène économique, l'eldorado européen. On continue à attirer les jeunes, fragilisés ou non d'ailleurs dans leur pays, ainsi que leurs familles, qui, souvent, les mandatent pour en faire des sources de revenus pour divers besoins dont ils estiment qu'ils seront Ce phénomène économique est adossé, cela a été dit également, à un phénomène mafieux évident. Nous connaissons bon nombre de filières ; monsieur le secrétaire d'État, nous pouvons même vous donner les tarifs par pays et par région dans ces pays, puisque ces éléments sont apparus dans les différents départements. Enfin, je vous le concède, monsieur le secrétaire d'État, l'évaluation de la minorité est un sujet extrêmement délicat, pour lequel il n'y a pas de réponse évidente. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, quand il est venu au congrès de l'ADF en octobre 2017, a pratiquement dit que cette mission d'accueil et d'évaluation devait relever de l'État. Ensuite, il a considéré que peut-être les départements pouvaient l'assurer pour le compte de l'État. Le problème, c'est que les moyens n'ont pas été au rendez-vous, loin de là,

qui est difficile à comprendre. À l'évidence, nous sommes confrontés à un état d'urgence qui est temporairement masqué par la crise sanitaire- on comprend bien qu'il est difficile de se déplacer en ce moment, vu la situation -, mais qui est appelé à prospérer, et nous ferions une erreur considérable en restant sur la même appréhension du problème après cette brève accalmie. Je pense qu'il faut nous mobiliser dès maintenant pour apporter des réponses qui soient plus solides que celles qui ont été les nôtres jusque-là. Enfin, dans cet état d'urgence, nous mettons en danger l'aide sociale à l'enfance elle-même dans les départements, notre capacité à l'assurer de façon satisfaisante, les départements eux-mêmes dans leurs finances, mais aussi les Français. Il a été fait état d'un certain nombre de faits délinquants, qui sont de plus en plus préoccupants, notamment dans les territoires d'outre-mer.